La séance est ouverte. Le compte-rendu intégral de la séance du mercredi 13 juillet a été publié sur notre site internet, nous n'avons pas reçu d'observation, y a-t-il des observations en séance. Je n'en vois pas. Le procès verbal et donc adopté. Madame la Ministre. Mes chers collègues. Mesdames et messieurs, chers famille qui était là, monsieur le maire de Sainte-Geneviève des Bois. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris, c'était le 2 février dernier la disparition de notre collègue Olivier Léonard, sénateur de l'Essonne et venait tout juste d'avoir Il nous a quittés à l'issue d'un combat long de plusieurs années la combat. Acharné contre la maladie. Il l'a menée avec courage et détermination. J'étais présent le très très belle cérémonie d'hommage organisée le 10 février à Sainte-Geneviève-des-Bois, à laquelle ont assisté de nombreuses personnalités politiques et j'allais dire, beaucoup d'habitants. Beaucoup d'habitants de Sainte-Geneviève et de l'Essonne. Au cours d'une intervention particulièrement émouvante, la présidente Laurence Rossignol il a relaté de manière très personnelle mais aussi pudique 35 années d'amitié indéfectible avec Olivier Léonard. Le président Jean-Claude Requier a aussi évoqué très justement les valeurs humanistes. Laïque et républicaine qu'Olivier Léonard avait en partage avec le groupe du Rassemblement démocratique social européen. La passion de l'engagement politique. Sans cesse guider l'avis d'Olivier Léonard c'était pour lui une manière de servir un idéal au bénéfice de l'intérêt général de ses concitoyens. Il était né le 29 janvier 1964 Suresnes dans une famille juive laïque. Ses grands-parents, nous l'avons évoqué avec la famille avait été victime du nazisme. Ce drame familial et sans doute à la racine, très profonde. Du combat permanent contre le racisme et l'antisémitisme, qui a été le sien et qu'il est bon de rappeler. à cet instant. à l'âge de 20 ans il fut en 1984 l'un des co-fondateurs de SOS Racisme, côté de Malek Bouti d'Harlem Désir et Julien Dray. Olivier Léonard s'était également engagé dans la vie militante en participant au mouvement des jeunes socialistes, et ce dès le début des années 80 à la veille de l'élection de François Mitterrand lorsqu'il était encore lycéen au lycée Turgot. Puis comme étudiant à la faculté de Tolbiac, des amitiés qui se sont poursuivies, bien au-delà de la faculté. Son engagement militant au sein de la gauche socialiste s'est poursuivi par la découverte du Parlement lorsqu'en 1991 il suivi à l'Assemblée nationale comme attachée parlementaire, Julien Dray, devenu député de l'Essonne. élu conseiller municipal de Geneviève des Bois en 1995 Olivier Léonard ont devint maire adjoint puis maire en 2001, s'investit à fond dans ce qu'il considérait être le plus beau des mandats et fut réélu maire à 2 reprises, en 2008 et 2014, preuve d'un réel attachement des jeunes au fait va à son égard. Il ne renoncera pas. Mais 22 2017 après son élection au Sénat, il dut se mettre en conformité avec la législation sur le cumul des mandats. Comme l'avait souligné, en février, notre collègue Laurence Rossignol, il s'était, je cite, révélé épanoui dans la fonction de maire, ce pourquoi il était fait. à l'occasion de son départ de la mairie, il exprimé avec beaucoup de justesse ce qu'incarne cette fonction, une passion pour l'intérêt général, l'amour de sa ville et aussi le dévouement total pour nos concitoyens dans tous les moments qui ponctuent leur quotidien, beaucoup d'entre nous qui ont connu cette vie de mère prenne dans les mots d'Olivier Léonard ce que ça veut dire réellement. Saison 2 mandats. Transforma sa ville, il la fasse a en quelque sorte à son image fait d'humanisme et de fraternité. Défenseur acharné de son territoire au sein de la grande couronne de l'Île de France, Olivier Léonard avait aussi compris que l'intercommunalité pouvait apporter une dimension supplémentaire à l'action publique, mais il a bataillé pour empêcher la constitution d'une intercommunalité géante, c'était la mode à l'époque de 800000 habitants et il a présidé à partir de 2008, une structure intercommunale à taille plus humaine d'ailleurs le nom vous l'évoquera la communauté d'agglomération du Val d'Orge, devenu en 2016 coeurs des sonne agglomération il y aura pour le développement d'activités économiques et culturels et d'emplois de proximité. Toujours et partout il appliqué le principe de Jean Jaurès, partir du réel pour aller vers l'idéal. Septembre 2017. Olivier Léonard si son entrée au Sénat. Il voyait dans le mandat parlementaire, une occasion de prolonger ses combats locaux notamment celui en faveur des départements de la grande couronne l'élu des Yvelines, que je suis n'est pas totalement indifférents à ce sujet, comme avec les autres collègues de l'Essonne qui étaient autour de moi ce jour là. Il voulait conforter la place et améliorer les conditions des habitants de la grande couronne. Olivier Léonard adhéra au groupe du Rassemblement démocratique et social européen et devint membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui a fait bénéficier de sa bonne connaissance des dossiers, notamment sur un sujet majeur pour lui, les transports. Il s'est notamment investi dans les travaux sur le projet de loi d'orientation des mobilités, le développement des mobilités était en effet l'un de ses chevaux de bataille, avec une attention particulière portée aux problématiques de desserte de proximité et de désenclavement géographique moyen de réduire les inégalités territoriales en 2020 et rejoignez la commission des affaires sociales, madame la présidente j'ai souvenir précis d'un entretien avec lui au sujet de l'égalité d'accès à la santé qui était pour lui essentiel si sa gratitude pour un système de soins qui l'accompagnait dans la solidarité et dans la qualité. Son état de santé ne lui permettait pas toujours de participer malheureusement autant qu'il aurait souhaité aux travaux du Sénat mais il tenait à venir siéger parmi nous dès qu'il le pouvez. Son combat. En faveur des Kurdes. à fait vibrer notre hémicycle 27 mars 2018, regardez le Journal officiel de nos débats, ce jour là. Il déclarait à l'occasion d'une question d'actualité, protéger les Kurdes, c'est défendre nos valeurs, c'est lutter contre le terrorisme, par conséquent, c'est aussi nous protéger nous-mêmes Dans la continuité de son action locale, il était aussi rester encore et toujours un inlassable défenseur de la laïcité lors d'un débat, c'est le 8 janvier 2020 Olivier Léonard s'exprime en ces termes : la laïcité, ce n'est pas un règlement ce n'est pas une loi, ce n'est pas un point d'équilibre, d'une manière sympathique de vivre ensemble, c'est la protection de tous les individus face à la tentation d'une norme philosophiques ou religieuses, promulguée hors de la démocratie, Représentant du Sénat au sein de l'Observatoire de la laïcité, à partir de février 2019 il s'appliqua fortement, là encore, comme toujours, on la défense des valeurs républicaines. Olivier Léonard a toujours eu pour ses concitoyens et ses administrés un exceptionnel dévouement. Je fais bien sûr référence à la tension permanente qu'il portait à chacun, mais je veux aussi souligner sa pudeur personnelle, son élégance morale, celui qui a toujours préféré une certaine discrétion à l'ostentation. Il était une référence d'engagement et d'altruisme savait aussi rassembler, fédérer autour de lui des personnalités venues d'horizons divers, au service des actions qu'il entreprenait et des valeurs qu'il défendait les valeurs pour lesquelles parfois ils savaient aussi cliver pour les affirmer avec force oui, mes chers collègues. Je souhaite que nous gardions d'Olivier Léonard le souvenir d'un sénateur à la fois chaleureux, un élu de proximité, profondément attachés à l'Essonne Sainte-Geneviève-des-Bois. L'image d'un humaniste de droiture, doté d'une culture étendue et d'une grande curiosité intellectuelle. à ses anciens collègues de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, ses collègues de la commission des affaires sociales à ses amis du groupe RDSE je voudrais redire tout le sentiment que nous éprouvons. à ses parents, Nelly et Gilbert. Qui sont en face de moi. à son épouse Nathalie, ces filles Lucie Laura et à Riom Frédéric son frère à sa famille, à ses proches, ses amis, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa vie, qui ont partagé ses engagements je souhaite redire comme je leur aux maires et aux élus de sa Geneviève des Bois en ce moment de de recueillement la part que le Sénat a pris réellement à leur deuil. Votre peine a été, et aujourd'hui encore la note nous avions noué ses Liens particuliers, les rester parmi nous, trop peu de temps, et pourtant il s'entend bien, en tous les cas pour ceux qui l'ont rencontré, qui ont partagé qui parfois se sont affrontés avec lui, ils ne sont pas indifférents au message d'Olivier Léonard il restera, ça n'est pas qu'un mot pourtant des loges présents dans dans nos mémoires et je dois dire que regardons. Le fauteuil qui était le sien à la fois les valeurs qui porte. Le Tricolore qui est aussi présent, les valeurs qui irradie quelque part, il est encore parmi nous. Madame la ministre, je vais vous donner la parole pour que vous vous exprimiez au nom du gouvernement, je donne donc la parole à Madame Isabelle Rome ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes chargés de la diversité et de l'égalité des chances des combats aussi qui a mené Olivier Léonard, Madame la Ministre. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, cher, membre de la famille d'Olivier Léonard monsieur le maire, il y a des discours que l'on prononce avec plus de gravité et de solennité que d'autres, celui-ci est de ceux-là, il y a des hommages qui nous plonge dans les coulisses de notre histoire contemporaine et des combats qu'elle charrie et celui-ci est de ceux-là, j'ai Olivier Léonard l'engagement au service des autres n'était pas un acquis. C'était inné, comme son amour pour la République et pour celle-ci, ce qui la peuplent l'engagement avec un E majuscule coulait dans ses veines, cette volonté de changer la vie des autres qui demeurera chez lui comme une seconde peau s'enracine dès 1980 alors qu'il n'est encore qu'élève au lycée Turgot, il adhère au Parti socialiste, la campagne de présidentielle de François Mitterrand le fascine, étudiant il s'arrime quelques années plus tard, un syndicat rocardien et le militant voit le jour, cette flamme ne se consume aura jamais. Une flamme dans l'incandescent jaillit à la, à la faveur de l'aventure, SOS Racisme avec ses compagnons de route de lutte, Julien Dray, Harlem Désir, notamment il redonne ses lettres de noblesse à 2 triptyque républicain de liberté, d'égalité et de fraternité, ils se battent alors pour suturer les plaies d'une société française disloqué une France plurielle dont il a voulu faire une République unie ces combats contre le racisme contre l'antisémitisme, contre la xénophobie, mais aussi contre l'extrême droite et les communautarismes seront au bout du compte, les combats de toute sa vie des combats qui se confondent avec l'universalisme républicain dont il fut un ardent partisan un infatigable défenseur. à l'aube du XXIe siècle, c'est le baptême électoral en 2001, il est élu à la tête de la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, ce mandat de maire auquel il était viscéralement t'attacher constituait pour lui une sorte de sacerdoce républicain en permanence au chevet et à l'écoute de ses administrés, Olivier Léonard ne comptait pas ses heures et ne me nageait pas son énergie 16 années durant son dévouement fut totale de sa commune, il a épousé tous les enjeux tous les atouts, tous les défis toutes les vicissitudes 16 années durant, il a ainsi embrasser toutes les joies et toutes les peines qui font le quotidien des maires de France, les Novès enfin qui lui ont renouvelé leur confiance, peuvent en témoigner l'action pour politique n'était pour lui, pas une fin en soi, ni un caprice et gothique, l'action politique, c'était au contraire cet idéal adolescent qui aspirait à changer la vie de nos concitoyens un idéal qu'une fois adulte, une fois j'ai lu, il n'a eu de cesse de rendre concret qu'il s'agisse de l'égalité des chances et du combat pour la méritocratie, qu'il s'agisse de désenclaver son territoire en militant, par exemple, pour améliorer la desserte du RER qu'il s'agisse de faire revivre un territoire à travers le projet d'aménagement de la base de 117 qu'il s'agisse. De promouvoir la laïcité, vous l'avez rappelé monsieur le président, partout et tout le temps et d'ériger des remparts face au poison qui les arts de la République, le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de haine et de communautarisme ou qu'il s'agisse aussi de défendre les populations kurdes car, selon lui, pour reprendre les mots de c'était pendant les juste la liberté est un bagne aussi longtemps qu'un seul homme est as servi sur la Terre. La vision qu'avait l'Olivier Léonard pour le Val d'Orge et pour notre pays se traduisait ton acte systématiquement d'une certaine manière, il avait fait sienne la Maxime de Bergson : agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Mesdames et messieurs les sénateurs, Olivier Léonard a rejoint les bancs de votre assemblée en 2017. Cette nouvelle écharpe de sénateur de l'Essonne n'a nullement émoussé l'intensité de ses engagements, bien au contraire, membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, puis à partir de 2020 de celle des Affaires sociales, il s'est notamment investi dans les travaux sur la loi d'orientation des mobilités, ainsi que sur celle de l'accès à la santé pour toutes et tous, changer la vie, encore et toujours, toujours à la proue du combat pour la défense de l'universalisme, vous l'aviez monsieur le président, nommé à l'Observatoire de la laïcité. Mesdames et messieurs les sénateurs, depuis 10 ans, ces combats d'élu local et de parlementaire que je viens sommairement de retracer Olivier Léonard les a mené de front avec un combat malheureusement plus intime, celui contre la maladie. Un combat sur lequel il avait je tiens à voile de pudeur qui l'a anobli d'une dignité supplémentaires, sa vie ne saurait être délié de ses engagements humanistes. à travers ces mille un combat Olivier Léonard n'a cessé d'offrir une voix et un visage à ceux qui en étaient privés, il n'a cessé de choisir le camp des plus fragiles, les opprimés des invisibles. Homme de gauche, sans pour autant s'enfermer dans les villes querelles politiciennes, il n'a cessé de s'opposer aux malheurs du monde. Parce qu'il ne supportait ni les inégalités ni la justice, et parce qu'ils conspuaient l'intolérance en d'autres termes, ne pas se mettre au service de ceux qui font l'histoire, mais de ceux qui la subissent, pour reprendre les mots prononcés par Camus à Stockholm un combat avec en sous-titre, une forme d'épée de Damoclès qui, chez lui, surplombe les tous les être s'humains. Ne sont jugés que sur leurs actes. En conclusion, permettez-moi d'avoir un mot. Pour son épouse Nathalie pour ses trois filles Lucie Laura Ariane et pour ses amis. Sachez que votre mari, votre père, votre ami. La si si une trace indélébile et qu'il gardera une place toute particulière dans la République, je vous remercie. Madame la Ministre, mes chers collègues. Mesdames et messieurs, chers famille. Je vous invite maintenant à partager un moment de recueillement à la mémoire d'Olivier Léonard.

Mes chers collègues, conformément à notre tradition en signe d'hommage à Olivier Léonard nous allons suspendre nos travaux pour quelques instants, si on s'donc suspendue, elle sera reprise à 15 heures 15 la séance est suspendue.

La séance est reprise. Monsieur le président du Sénat a reçu de Madame la première ministre communication du décret de monsieur le président de la République, en date du 13 juillet 2022 complétant le décret du 28 juin 2022 portant convocation du Parlement en session extraordinaire acte est donné de cette communication ce décret qui vous a été adressée, a été publié sur le site internet du Sénat. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne est parvenu à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle l'examen de 4 projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales pour ces 4 projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifiée, je vais donc les maîtres successivement aux voix. Je mais on voit le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord portant révision de l'accord général de coopération entre les États membres de la Commission de l'océan Indien. La commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption de ce texte. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il était adopté. Je mais aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention de coopération judiciaire internationale entre le gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations-Unies, représentée par le mécanisme international impartial et indépendant pour la Syrie. La commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption de ce texte qui est pour. Qui est contre qui s'abstient le projet de loi est adopté définitivement. Je mais on voit le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et l'Autorité bancaire européenne relatif au siège de l'Autorité bancaire européenne et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, la commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption, ce texte qui est pour. Qui est contre qui s'abstient le projet de loi est adopté définitivement. Je mais aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, la commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption, ce texte qui est pour. Qui est contre qui s'abstient le projet de loi est adopté définitivement. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'État du Qatar relatif au statut de leurs forces. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Olivier Becht Ministre délégué chargé du commerce extérieur de l'attractivité et des Français de l'étranger. Monsieur le président. Madame la rapporteure, mesdames et messieurs les sénateurs, je suis heureux et fier de présenter aujourd'hui le projet de loi visant à autoriser l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'État du Qatar relatif au statut de leurs forces, signé à Doha, le 24 novembre 2019 le Qatar constitue aujourd'hui pour la France un partenaire stratégique avec lequel elle a su nouer des partenariats aussi bien dans le domaine économique et culturel que dans celui de la Défense, la coopération militaire entre la France et le Qatar prend la forme d'activités de formation au profit des forces qatariennes et d'exercices conjoints dont certains sont assurés par des forces stationnées aux Émirats arabes unis, une vingtaine de militaires français sont par ailleurs déployés sur la base américaine d'Al-Udeid, dans le cadre de la lutte de la coalition internationale contre Daech. La coopération dans le domaine de l'armement est également significative le Qatar étant l'un des principaux importateurs d'armement français. En 2019, la France a pris l'engagement, en réponse à la demande des autorités qatariennes d'accompagner celle-ci dans l'organisation de la Coupe du monde de football 2022 afin d'en garantir la sécurité, la France déploiera des personnels et du matériel lors de cet événement et apportera son soutien au Qatar, dans le domaine de la sûreté aérienne et de la lutte anti-drônes afin de sécuriser juridiquement le déploiement de nos militaires appelés à se rendre au Qatar l'approbation du présent accord est indispensable, en effet, en l'absence d'accord relatif au statut des forces, le personnel français déployés sur le territoire qatariens seraient intégralement soumis au droit local sans bénéficier d'un statut de protection appropriée après plusieurs années de travaux et d'échanges avec le partenaire qatarien, il s'agit du premier accord relatif au statut des forces contenant une clause de partage de juridiction conforme à nos exigences constitutionnelles et conventionnelles signées avec un État du Golfe, il offre ainsi un cadre juridique protecteur à nos militaires rédigé sur la base de la réciprocité et s'inspirant des clauses classique figurant dans les accords du statut des forces, signée par la France, l'accord aujourd'hui soumis à votre examen détermine le statut juridique et et les conditions de séjour des personnels français déployés au Qatar et des personnels qatarien déplorait en France dans le cadre d'activité de coopération en matière de défense, les membres du personnel ainsi que les personnes à leur charge, sont tenus au respect de la législation de la partie d'accueil, c'est bien normal, ils sont autorisés à pénétrer sur le territoire de la partie d'accueil et a quitté celui-ci a, sous réserve de détenir un passeport et un VISA et moyennant la communication préalable de leur identité aux autorités de la partie d'accueil en matière de dépenses la partie d'envoi paye les frais occasionnés par ses activités dans l'état d'accueil en cas de nécessité ou d'urgence, les actes médicaux, de même que les évacuations sont effectués à titre gratuit en matière fiscale, la domiciliation des membres du personnel et des membres de leur famille, dont ils ont la charge est maintenu dans l'état d'envoi en outre la partie d'envoi peut importer et réexporter en franchise de droits de douane et de taxes, les matériels destinés à l'usage exclusif de ses forces sur le territoire de la partie d'accueil en matière pénale, l'accord prévoit un partage de juridiction les infractions commises par un membre du personnel de la partie d'envoi ou par une personne à sa charge relève en principe de la compétence des juridictions de la partie d'accueil cette compétence est toutefois dévolu prioritairement aux autorités compétentes de la partie d'envoi lorsque l'infraction a été accompli dans le cadre du service ou lorsqu'il a été porté atteinte aux biens ou à la sécurité de la seule partie d'envoi et ou du personnel de celle-ci, en cas de poursuite devant les juridictions de la partie d'accueil, la personne concernée bénéficie des garanties du droit à un procès équitable, et en particulier du droit à être jugé dans un délai raisonnable et être représenté ou assisté à bénéficier d'un interprète à communiquer avec un représentant de son ambassade à être informé des accusations portées contre elle et à ne pas se voir appliquer de rétroactivité de la loi pénale. Si les poursuites intentées aboutisse à une condamnation dans l'état d'accueil, l'accord prévoit que ce dernier examinera avec bienveillance les demandes tendant à permettre à la personne condamnée de purger sa peine dans l'état d'envoi

l'autre État, ce dernier ne remettra au premières état une personne faisant l'objet de poursuites que contre l'assurance que ces peines ne seront ni requise, ni prononcée ou si elles sont prononcées qu'elles ne seront pas exécutées, la peine de mort étant toujours en vigueur, au Qatar, la France a inséré dans l'accord, cette clause de juridiction conforme à nos exigences constitutionnelles et conventionnelles, résultant notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il était essentiel pour la France que l'accord écarte toute possibilité d'application de la peine de mort ou d'un traitement inhumain et dégradant, qu'un : pour un Français ayant commis une infraction au Qatar que pour 1 qatarien ayant commis une infraction en France et dont le Qatar demanderaient la remise les garanties que la France a obtenu dans cet accord sont absolument explicites sur ce point fondamental : telles sont, monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'État du Qatar relatif au statut de leurs forces, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposer à votre approbation, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sylvie gouache avant, rapporteur de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour dix minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant de revenir sur les principales stipulations de cet accord. Je dirais, quelques mots sur les relations qu'entretient la France avec le Qatar afin de mieux appréhender l'intérêt de ce texte et le contexte dans lequel il s'inscrit. Le Qatar est un allié stratégique de la France dans un contexte de fortes tensions au Proche et Moyen-Orient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Levant, le pays accueille 24 personnel de notre armée de l'air et de l'espace engagés dans l'opération Chammal est déployée sur la base militaire américaine d'Al-Udeid. Par ailleurs, au Sahel, le Qatar a fourni un appui capacitaire, à la force conjointe du G5 Sahel en livrant une cinquantaine de véhicules blindés au Mali et au Burkina Faso, le partenariat franco-qatarien s'exprime aussi dans le domaine industriel de défense, d'après le dernier rapport au Parlement sur les exportations d'armement de la France, le Qatar était le 1er client de la France pour la période de 2015, 2020 avec près de 18 pour 100 des commandes d'armes françaises ces dernières années, le pays a notamment signé de contrat pour la quitter l'acquisition de 36 Rafale au total qui pour l'essentiel, ont déjà été livrés. Compte tenu de ces grands contrats d'armement, le le notre coopération militaire prend également la forme d'activités de formation au bénéfice des forces armées qatarienne ainsi ces dernières années, quelque 230 qatariens ont été formés au pilotage du Rafale sur la base aérienne de Mont-de-Marsan et une quarantaine de personnel a suivi des études dans nos écoles militaires. Enfin, lors de la crise afghane d'août 2021, le Qatar a appuyé la France dans l'opération Apagan opération d'évacuation de ressortissants français et afghans, ces derniers étaient pour la plupart d'anciens auxiliaires de l'armée française menacée en raison de leur engagement aux côtés de notre pays. J'en viens à présent au contenu de l'accord. Son objet est de renforcer le cadre juridique de notre coopération militaire avec le Qatar en définissant les principes de sa mise en oeuvre. L'absence d'un tel accord constitue aujourd'hui un réel frein à l'approfondissement de nos, de nos relations bilatérales en ce domaine, à titre d'exemple, le plan annuel de coopération franco-qatarien comprend une centaine d'actions mais moins de la moitié, a pu être mis en oeuvre faute d'instruments juridiques couvrant l'intégralité des champs de la coopération. Les dispositions de ces accords s'appliqueront tant au personnel militaire qu'aux personnels civils, par exemple, les agents de la direction générale de l'armement, appelés à se déplacer dans le cadre des contrats d'armement. Le texte soumis à notre examen et de factures tout à fait classique il régit notamment les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre partie, le port de l'uniforme et des insignes militaires ainsi que la détention le port et l'utilisation des armes de dotations par les militaires de chaque parti. En outre, les parties reconnaissent sur leur territoire la validité des permis de conduire pour les véhicules et engins militaires de l'autre partie. Enfin, il est important de souligner que cet accord est conforme à nos exigences constitutionnelles et conventionnelles, comme l'a dit Monsieur le Ministre, il s'agissait d'une condition sine qua none à sa signature puisque le Qatar continue d'appliquer la peine capitale en effet en 2020 ressortissants népalais a été exécuté à la suite de sa condamnation à mort pour meurtre, ce qui a mis fin au moratoire observé dans le pays depuis 2003. L'article 11 de l'accord franco-qatarien protège ainsi les membres du personnel et les personnes à charge des 2 États. Contre la peine capitale et les traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces peines ne seront ni ni remise ni requise, ni prononcée, si toutefois elles étaient prononcées ne serait alors pas exécuté, il convient de souligner à cet égard que les termes de cet accord protège à la fois les personnels français et les personnes à leur charge, mais également les personnels qatarien soumis à la juridiction française et pouvant faire l'objet d'une mesure d'extradition ou d'expulsion. Cet accord répond donc aux intérêts de la France en ce qu'il renforce le cadre juridique de notre partenariat noué dans une région stratégique pour notre défense et pour notre sécurité. Il vise à définir le statut juridique des personnels civils et militaires du ministère des Armées lorsqu'ils sont amenés à se rendre au Qatar pour une opération extérieure ou une activité de coopération. L'adoption d'un tel texte n'est évidemment pas un blanc-seing donné au gouvernement ou à l'État, du Qatar, ce partenariat peut susciter des interrogations légitimes. S'agissant notamment du respect des droits de l'homme dans ce pays, mais le but de cet accord est précisément de protéger les ressortissants français qui se rendent dans l'émirat pour mettre en oeuvre cette coopération. sais que mes chers collègues, soyons pragmatiques, quelle que soit l'issue du vote, la coopération franco-qatarienne continuera d'exister, et même de se renforcer en effet le sénat ne se prononce pas aujourd'hui sur la nature des Liens tissés entre la France et le Qatar, dans le domaine de la défense mais bien sûr l'accord relatif au statut de nos forces. Le Parlement n'est pas non plus consultés sur la question des exportations d'armement, ce que l'on peut regretter, Monsieur le Ministre, en effet, malgré un timide, renforcement de l'information au Parlement sur le sujet, les représentants de la nation reste exclu des processus de décision et de contrôle, car nous nous sommes, nous ne sommes consultés ni a priori, c'est-à-dire sur l'attribution des licences d'exportation par la Commission interministérielle pour l'étude des exportations, des matériels de guerre ni a posteriori dans le cadre du contrôle assuré par un comité ministériel ad-hoc. Voilà pour conclure, mes chers collègues, je vous invite donc à adopter ce projet de loi, comme l'a fait, la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées du Sénat, en février dernier, je vous remercie. merci, madame la rapporteure de la. Suite de la discussion générale, la parole est à monsieur rendrez guignol pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission madame le rapporteur, mes chers collègues, le développement d'il y tôt le Qatar et la France n'est plus à démontrer depuis longtemps nos 2 pays, échange de nombreux dans de nombreux secteurs, notre collègue rapporteur a très bien exposé dans le contexte actuel de la crise avec la Russie, j'insisterai tout d'abord sur la nécessité de densifier encore davantage nos échanges dans le domaine de l'énergie à cet égard, je me réjouis de la sélection par le gouvernement qatari de Total énergies comme 1er partenaire de projet INF, eux, une décision qui permettra d'augmenter la capacité d'export du GNL bas-carbone vers l'Europe. Comme la presse précédemment souligné le commissaire européen Marché intérieur Thierry Thierry Breton, un grand projet de gazoduc euro-arabe tracerait les perspectives de moyen et long terme en matière de sécurité des approvisionnements cette filière constitue aujourd'hui une réponse certes partielle au défi du changement climatique et de la transition énergétique à laquelle nous devons répondre et devrait atténuer la tentation de réouverture des centrales à charbon constater ici et là, s'agissant des questions de sécurité de défense qui focalise déjà une grande partie des échanges entre Doha et Paris, elles doivent bien entendu être approfondie de déclarations d'intention relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment à celle relative à la mise en place de dialogue stratégique de nombreux outils renforce régulièrement notre relation bilatérale d'une relation qui contribue à la sécurité globale pour le RDSE, c'est une bonne chose, compte tenu de la situation sécuritaire du Proche et Moyen-Orient. Je n'oublie pas l'appui fourni par le Qatar à la force conjointe du G7 G5 Sahel ou encore son implication dans l'opération Apagan dans le quart de la crise afghane un Cadre de confiance et de coopération militaire c'est ainsi durablement installée entre la France et le Qatar depuis cela implique et d'ailleurs plus que nos forces, j'en viens ici à nos projets de loi sur le statut des forces, bien que ce texte soit indépendante des événements de la Coupe du monde de football qui se profile, sans se prononcer sur l'opportunité d'une telle compétition dans un pays plus connu pour les richesses de son sous-sol que pour ses pelouses se qui se profile, nous avons tout intérêt à adopter rapidement car constitue un gage de bonnes intentions de la part du Qatar aux relations de nous nos exigences constitutionnelles et conventionnelles, ça a été dit, pour autant, nous savons pourquoi ce texte est sorti de la procédure d'examen simplifiée en mai 2020, l'exécution de ressortissants n'est pas les condamnés à mort par la justice qatarie inquiète légitimement qui est devenu le moratoire sur les exécutions de mise en place depuis 2003. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, dans la droite ligne de votre prédécesseur, Jean-Yves Le Drian, le développement de nos relations avec le Qatar ne doit pas empêcher la tenue d'un dialogue positif lucide et exigeant, d'autant que la fermeté peut porter ses fruits, on a pu le constater concernant le droit du travail, la pression de porter sur Doha par de nombreux pays occidentaux dont le nôtre, a permis d'améliorer une situation dramatique et scandaleuse dans le secteur du bâtiment, certes, tout n'est pas à la hauteur de nos attentes, mais de tels accords comme celui dont il est question aujourd'hui contribue à converger vers un minimum de standard car ou de la protection de nos ressortissants concernés par cet accord, c'est aussi par la multiplication de ce type de relation entre pays, au demeurant très différent que les progrès sensible hein, le domaine des droits de l'homme peut être acté, c'est pourquoi le groupe mon groupe approuvera ce projet de loi, je vous remercie. Merci, cher collègue, dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Michael pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour six minutes. Sous le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, rapporteurs, mes chers collègues. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui et qui a été adopté par nos collègues députés pour technique ou formelle qu'il puisse paraître ne saurait être examinée ainsi que j'avais pu l'exprimer à cette même tribune à propos de l'accord similaire relatif à l'organisation de la prochaine Coupe du monde de football au Qatar en nous contentant d'une simple étude de texte et sans nous interroger sur le contexte sur le texte et ses effets juridiques, le propos est assez simple : ça a été rappelé à plusieurs reprises là. France et le Qatar ont établi de longue date un partenariat militaire stratégique, cette relation privilégiée se traduit concrètement par la vente, par exemple, d'avions de combat l'armée de l'air qatariennes et par la formation de ses pilotes de chasse, on notera que sur la décennie 2010 2020, le Qatar et tout de même le 2ème, client de la France en matière d'armement, sans compter les autres achats que le Qatar effectue. Auprès de pays européens, on voudrait que certains pays européens, eux-mêmes en fassent autant, quand il décide de se réarmer de manière conséquente, j'ajoute à cela, ça a été rappelé par Madame la rapporteure l'aide du Qatar dans l'évacuation des ressortissants d'Afghanistan et tout un ensemble d'autres apports dans cette. Coopération, mais ce partenariat stratégique va bien, nous, de la, de ses seuls aspects commerciaux, nos 2 pays organisent régulièrement des exercices militaires et la France a pu compter sur le soutien des forces amies qatariennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamique au Sahel et au Levant, l'approfondissement de ce partenariat, impose une convention bilatérale protégeant les droits et libertés fondamentales de nos forces de l'ordre lorsque celles-ci se trouvent en territoire qatarien la sur lequel nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui répond à cet impératif puisque, ainsi que l'ont rappelé monsieur le ministre et Madame la rapporteure, si les forces de l'Ordre sont tenus de respecter la législation qatarienne, celles-ci ne peuvent être privés du droit hein. Procès équitable et ne peuvent encourir la peine de mort, mais mes chers collègues, je l'ai déjà expliqué lors de l'examen sur le texte sur la Coupe du monde donc, bis répétita autour du texte, il y a le contexte et se pose la question de la crédibilité de la France dans le choix de ces coopérations militaire, voilà une question précise qui appelle une réponse claire car chacun le sait, il faut aller vers l'Orient compliqué avec des idées simples, alors disons les choses simplement les droits et les libertés fondamentales pour lesquelles la France a payer. Un lourd tribut au cours de son histoire, sont régulièrement bafoués par le Qatar, la Coupe du monde, dites de la honte dans les conditions d'attribution sont entachés de soupçons de corruption amène une lumière crue sur la réalité de l'état de droit dans l'émirat et interroge sur l'opportunité d'un tel niveau de coopération et sur sa signification politique, il convient de rappeler à cette tribune que le processus d'attribution de l'événement fait en ce moment même l'objet de procédures judiciaires lourdes, les magistrats du parquet national financier ont ouvert une information judiciaire pour corruption et pour recel et blanchiment des procédures similaires ont actuellement cours aux États-Unis et en Suisse, et c'est à très haut niveau, que ces faits de corruption sont présumés dans l'entourage des plus illustres supporters français du Paris Saint-Germain qatarien interroge également et même scandalise les conditions de travail épouvantables, des milliers de travailleurs étrangers sur les chantiers de construction des stades. Pas un de nous ici ne pourrait les supporter plus de 48 heures, quand je dis 48 heures je suis large si l'Organisation internationale du travail, et plusieurs ONG salut certaines avancées, comme l'ouverture récente d'un bureau de l'Organisation internationale du travail ou l'abolition de la kafala nombreuses sont les organisations de défense des droits de l'homme, qui continue de les trouver profondément insuffisantes et qui mettent en doute le nombres de ce qu'on appelle formellement les morts au travail et c'est dans une perspective internationaliste, nous semble-t-il, que doivent toujours tu es toujours être défendue, les conditions de travail des ouvriers j'ajoute pour terminer que construire des stades climatisés, lorsque l'on est dans le peloton de tête mondiale des pays producteurs de carbone, c'est-à-dire statistiquement 6 fois plus que la Chine par habitant ne vient pas rehausser le le tableau. Vous avez parlé Madame la rapporteure d'interrogations légitimes et elles existent, comme je viens de les exposer, il est donc aisé de comprendre qu'au regard du décalage constaté entre cet accord de coopération, accepté par le gouvernement et la réalité de l'État droit au Qatar, donc trop groupe ne pourra voter ce texte, seule la protection offerte. à nos forces de l'ordre protection nécessaires. Nous empêche de voter contre, nous ne nous l'interdisons que pour elle et pour elle seule, en conséquence, le groupe socialiste s'abstiendra. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Abdallah Hassani pour le groupe RDPI pour ce 4 minutes.

Cet accord, qui est le fruit de 5 années de négociations comportent des vraies avancées. Il offre un cadre juridique protecteur à nos personnels français déployés au Qatar et à leurs proches qui les accompagne jusqu'ici soumis aux lois qatariennes et notamment à la peine de mort qui, rappelons-le, est toujours en vigueur, au Qatar, ça a été dit tout à l'heure si le retour à la procédure normale de l'examen de ce projet de loi peut être l'occasion de dresser un état des lieux de notre relation bilatérale avec le Qatar, il ne doit pas se transformer, mais semble-t-il en procès à l'endroit de cet état. Ce serait vain et stérile. L'examen de cet accord advient dans un contexte. Aussi inédite qu'à certains, à raison de la guerre en Ukraine et c'est en temps de crise qui les partenariats stratégiques que la qualité des relations bilatérales prennent tout leur sens, la crise afghane, un autre 2021 Anne, elle est un exemple signifiant, c'est avec l'aide active du Qatar qui nous avons pu exfiltrer vers doit plus de 300 français et afghans, preuve de l'importance de la qualité de cette relation bilatérale, dans une région historiquement instable, il est vrai néanmoins que nos relations avec le Qatar ne doivent pas occulter les sujets de discorde tels que le respect des droits humains, la condition des femmes et la protection des travailleurs étrangers, nous devons en ce domaine, rester lucide vigilants, exigeants, le fait dans la presse internationale se fait l'écho interroges certes nos consciences mais il ne saurait occulter les progrès faits par le Qatar, que ce soit en termes de droits sociaux, des droits des femmes ou des salaires minimum, les femmes occupent désormais au Qatar, des postes de responsabilité dans de nombreux secteurs, à titre d'exemple, plusieurs femmes sont ministre actuellement le Qatar a été le 1er pays de la région à abroger le système de la kafala système de mise sous tutelle étroite de tout travailleur étranger si l'indéniable OK, du chemin reste à parcourir, comparé aux standards français en matière de démocratie et d'état de droit, des progrès tangibles sont réalisés en somme parce que cet accord renforce le cadre juridique de la relation bilatérale de défense avec le Qatar, dans un contexte de tensions croissantes dans le Golfe arabo-persique et au-delà, le groupe RDPI votera ce projet merci. Merci, cher collègue, dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Emmanuel Capus pour le groupe, les indépendants pour cinq minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La semaine dernière l'examen en commission des affaires étrangères de divers projets de loi approuvant des conventions internationales n'a suscité aucune opposition. Le groupe écologiste a cependant souhaité que nous en séance publique de celle conclue entre la France et le Qatar, cette convention vise à préciser le statut des forces armées déployées réciproquement dans ces 2 États, et concernent notamment le partenariat liant la gendarmerie nationale et la force qatarienne de sécurité intérieure. Le Qatar et la France coopère sur de nouveaux sujets, éducation, culture, mais aussi économique, notre coopération se développe également dans le domaine sécuritaire, le Qatar, apprécie l'expertise française en la matière, déployés notamment dans le corps de l'exercice Golfe Falcon. La France et son partenaire ont en outre initiée en 2019 un dialogue stratégique, le Qatar est par ailleurs l'un des principaux acquéreurs de l'armement français, il a ainsi commandé 36 avions Rafale dans les 7 dernières années. Certains s'émeuvent parfois du fait que la France figure parmi les 3 plus grands exportateurs mondiaux, c'est pourtant la condition de notre souveraineté, la seule commande de nos armées ne pourrait suffire à la viabilité de notre industrie de défense, l'export est essentiel à notre souveraineté. Le Qatar a par ailleurs maintes fois démontré son attachement à la recherche de solutions négociées aux divers conflits que qu'on ait la région, ce fut le cas lors de l'accord de Doha en 2015. Son retrait en 2017 de la coalition menée par l'Arabie Saoudite lui permet également de faciliter le dialogue dans la guerre au Yémen, c'est le Qatar encore qui a proposé son aide pour débloquer les négociations sur le nucléaire iranien. Le partenariat noué entre la France et le Qatar et bénéfique pour nos 2 États notre relation privilégiée, a ainsi été particulièrement précieux au mois d'août dernier, lorsqu'il s'est agi texte filtrer en urgence nos personnels de l'Afghanistan. Le Qatar a également participé à l'opération Barkhane. Cette relation de coopération sert dont nos intérêts mais le permet également de diffuser nos valeurs. Nous voulons croire que la relation de la France à contribuer à l'amélioration relative des droits de l'homme au Qatar. Le droit du travail, a connu de nombreuses avancées depuis 2020 les employeurs ne peuvent plus détenir les passeports de leurs employées, l'exigence d'un VISA pour quitter le territoire a été supprimé et un salaire minimum est désormais en vigueur. La condition de la femme a également connu des progrès, elle bénéficie ainsi de plus de liberté que dans bon nombres des États de la région, que ce soit en matière d'habillement d'éducation ou encore de travail. C'est au Qatar, que les femmes sont les plus présentes sur le marché de l'emploi. fini ne signifie pas pour autant que ce jeune pays qui progresse vers la démocratie, partage, j'avais le monde des valeurs identiques comme on nous avions eu l'occasion de le dire lors du texte portant sur la sécurité de la Coupe du monde 2022, c'est par la coopération que nous pourrons amener nos partenaires à se rapprocher de nos valeurs de tolérance et de liberté. Quelles que soient les difficultés, l'indignation ne suffit pas. La France occupe une place bien particulière dans le monde et elle constitue une source d'inspiration pour nombres de pays. Les membres du groupe, les indépendants sont convaincus que son action dans le monde si elle implique, comme toute action une forme de pragmatisme permet de diffuser et de renforcer nos valeurs.

Monsieur le président, monsieur le président de la Commission, monsieur le Ministre, mes chers collègues, ouverte au lendemain de l'indépendance du Qatar, les relations diplomatiques, que la France entretient avec Doha célèbrent cette année leur 50ème anniversaire au fil de ce demi-siècle, la coopération bilatérale qui lie nos 2 pays n'a cessé de se renforcer et s'est notablement accélérée ces dernières années pour faire de ce petit pays du Golfe, un partenaire incontournable de la France dans la région particulièrement dense, nos relations se déploie dans le domaine économique, sportif, culturel et universitaire, mais aussi et c'est celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui dans le domaine militaire, bien entendu, le Qatar est un client très important de l'industrie française de l'armement, le deuxième sur décennies passées avec en particulier de nombreuses commandes dans le secteur aéronautique, c'est une donnée tout à fait majeur mais l'autre coopération militaire qui se font notamment sur l'accord de défense signé en 1994 s'avère plus profonde et ne se limite pas aux seules ventes d'équipements aux activités de formation qui en découlent, elle se traduit également au niveau opérationnel, notamment par la présence d'officiers français au sein de l'État-Major qatarien et par la conduite régulière d'exercices conjoints, c'est en outre déployé c'est bien année en lien avec des tables d'opérations majeure pour la France comme le Sahel, l'Irak ou la Syrie je tiens par ailleurs à saluer le rôle joué plus récemment encore par les autorités qatariennes pour faciliter la mise en oeuvre des opérations d'évacuation de nos compatriotes, mais aussi de nombreux citoyens afghans lors de la chute de Kaboul, la position stratégique du Qatar au coeur du Golfe arabo-persique, l'importance de ses ressources énergétiques, la diversification et son influence économique croissant les partenariats qu'il a su nouer avec des acteurs, des acteurs aussi nombreux que différents ses rapports, désormais en voie de normalisation avec ses voisins immédiats, sa volonté manifeste nous tout le monde, tous ces éléments plaident t'en faveur d'une consolidation de la relation déjà forte que nous entretenons avec cet État clé du Moyen-Orient, l'accord sur le statut des forces qui nous est soumis aujourd'hui il concourt épouse un nouveau jalon dans notre coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité car, en définissant de manière détaillée le droit applicable au personnel français des prix sur le sol du Qatar et réciproquement, il fournit dans de nombreux domaines très concret, un cadre juridique clair et pérenne à même de faciliter et donc de stimuler notre Colbert Haution opérationnel surtout il battu un cadre plus protecteur pour nos militaires et leurs familles par rapport à l'heure à la situation actuelle, qui ne prévoit pas qu'un régime particulier juridique puisse leur être appliquée, ce qui inclut une Exposition à la peine de mort, toujours en vigueur, au Qatar, certes, il existe depuis 2003 un moratoire qui rend, en théorie inapplicable, recours à la peine capitale, mais outre le fait que celui-ci a connu une entorse en 2020 il était néanmoins fondamental que l'accord conclu de 24 novembre 2019 contiennent une disposition permettant de protéger nos ressortissants contre ce risque pour des raisons de principes et de sécurité bien sûr mais aussi de sérénité pour les hommes et des femmes dont la présence secrétaire est lié d'une manière ou d'une autre au service de la France, au-delà de cette clause particulière, le reste de l'accord est de nature relativement générique, il apparaît semblable aux nombreuses autres textes de cette nature, plus de 80 à ce jour signé par la France avec d'autres pays, sa conclusion est néanmoins rendue particulièrement nécessaire dans le contexte de la prochaine Coupe du monde de football, en effet, la France s'est engagée à contribuer de manière significative à sa sécurisation et envisage pour ce faire, de mobiliser sur place davantage de personnel qu'à l'accoutumée, au-delà des divers questionnements qui peuvent entourer l'organisation de ce grand événement au Qatar, il était donc important que la sécurité juridique la plus robuste possible puisse être apportée à nos compatriotes dans l'exécution de leur mission reste bien sûr la question fondamentale des droits de l'homme, si elle n'a pas de lien Direct avec le texte que nous aime, examinons aujourd'hui elle suscite néanmoins de légitimes interrogations car personne ne peut il nous ignorer le Qatar demeure à ce jour très éloigné des standards que la France promeut en la matière, je note toutefois que par rapport à d'autres pays de la région, il a connu des avancées encourageantes, qu'il s'agisse par exemple des droits des travailleurs étrangers et des droits des femmes, je conviens naturellement que dans ces domaines comme dans bien d'autres, les progrès qui restent à accomplir son énorme, je ne me berce pas non plus d'illusion en imaginant que le Qatar comme d'ailleurs ses voisins pourraient du jour au lendemain, adoptée le socle de valeurs qui le socle ce cheminement sera nécessairement long et sans doute sinueux, je me félicite néanmoins que nous puissions en constater les prémices au sein de la société qatarienne, en outre, il me semble, en ce domaine, la voie du dialogue, un dialogue certes exigeant, il est toujours préférable à celle de l'ostracisme, c'est je crois la méthode la plus efficace pour accompagner ces évolutions positives qui ont eu lieu ces dernières années, et pourquoi pas, ont suscité de nouvelles pour l'ensemble de ces raisons, le groupe, les républicains se prononcera donc en faveur de la promotion de cet accord qui m'apparaît tout à la fois conforme aux intérêts de la France, il y a ceux de nos personnels amenés à la servir sur le territoire qatarien je vous remercie. Merci, cher collègue. à la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Guillaume Gontard pour le groupe écologiste solidarité territoire pour 4 minutes.

comme nous l'avions fait pour l'accord établissement un partenariat pour la sécurité de la Coupe du monde 2022 avec le groupe écologiste solidarité et territoires, nous avons demandé le retour à la procédure normale pour ce projet d'accord entre la France et le Qatar relatifs à l'état de nos forces, d'une manière générale, nous nous étonnons, et nous nous inquiétons que les Liens politiques, diplomatiques, militaires, économiques qui lient notre République avec la monarchie qatarie ne fasse l'objet de presqu'aucun débat au sein de notre classe politique le Qatar est pourtant loin d'être un partenaire comme les autres, rares sont les pays au monde qui respecte aussi peu, ça a été rappelé les droits humains les plus fondamentaux plus rares encore sont parmi ces pays, ceux avec lesquels nous entretenons une relation aussi étroite et aussi peu exigeante, alors que nous entamons un nouveau mandat, il nous paraît essentiel d'avoir ce débat dans notre hémicycle et pour savoir notamment si Monsieur le Ministre vous infléchirait quelque peu la position française des 5 dernières années, ce texte ambitionnant de renforcer la sécurité juridique pour les citoyens français au 1er rang desquels nos militaires et des citoyens qataris en France n'est pas la convention la plus problématique qui nous est soumise, elle est beaucoup moins que notre participation déshonorante à la sécurité de la Coupe du monde de la honte que nous avons vivement condamné en février, mais ce n'est pas un simple texte qui permettrait de sécuriser la présence de militaires français au Qatar ou de militaires qataris en France, il va plus loin qu'une simple sécurité juridique et représente une Pierre supplémentaire de la relation étroite que nous construisons avec l'émirat. Bon, nous nous interrogeons le bien-fondé et dont nous condamnons l'étroitesse parfois complice, fort de la respectabilité internationale qui lui confère l'organisation d'un événement planétaire, l'émirat se permet, par la voie d'un responsable de la sécurité de la Coupe du monde de sommer les sous les supporters LGBTQ il a plus qui se rendront à la Coupe du monde de se tenir à carreau, pire encore, la presse est venu mettre en lumière les dispositions légales qatari qui condamne à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison les relations sexuelles hors mariage et les relations homosexuelles, or l'article 11 de la présente convention stipule que la partie d'accueil exercé exerce par priorité son droit de Rugy de juridiction, nous allons donc soumettre nos soldats, nos soldats et nos soldats assez lois et assez peines incompatible avec le respect le plus Blazic des droits humains. Soulagement tout de même les alinéas 11 8 et 11 9 protège les membres du personnel et les personnes à charge des 2 États contre la peine de mort, toujours en vigueur au Qatar et contre les traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tenter de nous rassurer : le rapport de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale faisait preuve d'un manque d'exhaustivité qui confiné à la partialité et a été dénoncée comme telle, notamment par notre estimé ancienne collègue Marie-George Buffet, celui de la commission du Sénat en version sa fille n'est pas non plus à la hauteur de la responsabilité qu'induit le renforcement d'un tel partenariat si la France souhaite établir avec le Qatar, un dialogue lucide et et exigeant sur les droits humains, ce n'est certainement pas en fermant les yeux sur les châtiments corporels, la soumission des femmes, les discriminations ou encore les conditions de travail ayant entraîné la mort, ça été rappelé de près de 6500 ouvriers esclaves sur les chantiers de la Coupe du monde pour toutes ces raisons, pour la dynamique global dans lequel il s'inscrit le groupe écologiste votera contre cet accord et au delà, réitère son appel au boycott diplomatique de la Coupe du monde 2022, même en période de crise énergétique tous les reniements ne sont pas autorisés merci. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Pierre Laurent pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour 4 minutes. merci. relatif au statut de leurs forces armées dans cet accord figure un certain nombre de clauses visant notamment à sécuriser juridiquement les ressortissants français sur place, face, notamment, comme cela a été rappelé à la peine de mort ou à des traitements inhumains et dégradants mesure toujours appliquée par la justice féodale qatari c'est dire d'emblée la haute estime dans laquelle nous tenons la justice de ce pays pour de voir adopter une telle un tel statut, ce qui ne nous empêche pas, ou en tout cas, certains d'entre nous de continuer à qualifier le Qatar de partenaires stratégiques, comme l'avait souligné nos collègues députés communistes à l'Assemblée nationale, cet accord n'est du coup pas un simple texte technique, il s'inscrit de fait dans une collaboration étroite entre les forces armées françaises et qatari dans la continuité de notre alliance avec ce pays ainsi ces dernières années, pour ne citer que cet exemple, quelque 234 Arion étaient formés sur l'avion Rafale sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, la relation de la République française au Qatar, doit pour le moins pourtant nous interroger au Qatar, même si quelques mesurettes ont été prises récemment sur les les la situation reste proprement catastrophique et inhumaine du point de vue du respect des droits, en particulier pour les femmes et pour les millions de travailleurs étrangers de ce pays, je rappelle que les travailleurs étrangers au Qatar, c'est 80 % de la population du Qatar, si la situation des travailleurs étrangers s'améliore donc un tout petit peu, par exemple, avec l'autorisation de changer d'emploi, ces travailleurs sont soumis à des conditions qui sont qualifiés par toutes les associations de droits humains de travail forcé, ils sont payés dans l'écrasante majorité des cas au lance- pierres, sur la base de contrats que l'employeur ne respectent pas, quand ils existent, dans un pays dépourvu quasiment de tout droit au travail et où les syndicats et les partis sont de fait interdits, cette situation a été révélé au grand jour à l'occasion des chantiers de la prochaine Coupe du monde de football, on parle de plusieurs milliers de morts sur les chantiers personne désormais ne peut faire comme s'il n'était pas au courant, par ailleurs, ce texte sincère dans une coopération militaire qui tend à se développer et à d'importantes exportations de matériels français militaire vers le Qatar, comme cela a été rappelé en commission, d'après le 1er rapport au Parlement sur le sujet, le Qatar était le 3ème, client de la France pour la période 2016, 2020 avec 18 % de commande d'armes françaises ces dernières années, le pays a notamment signé de contrat pour l'acquisition de 36 Rafale, or cette relation militaire comme celle que nous entretenons avec les autres pétromonarchies du Golfe pose de graves problèmes ces pays qui vivent de rentes pétrolières sans avenir et méprisent les droits humains peuvent-ils être réellement des alliés stratégiques stable et durable pour la France, d'autant qu'ils usent tous, à commencer par le Qatar Doral de relation trouble dans les zones de guerre et de relations troubles avec les forces djihadistes à ce sujet, permettez-moi de rappeler que de à Doha a accueilli pendant des années, pendant la guerre en Afghanistan la représentation politique des talibans, c'est d'ailleurs de ce pays le 17 août 2021 alors que les États-Unis se retirent d'Afghanistan qu'à bord d'un avion militaire qatari, le Mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur des talibans, numéro 2 de ce mouvement, a rejoint la ville de Kandahar et fait son grand retour dans le pays, vous comprendrez donc que sans être opposé évidemment aux dispositions de protection juridique de cet accord pour les ressortissants français, nous considérons que ce texte s'inscrit directement dans une relation toxique de la France avec le Qatar, c'est en ce sens que nous nous y opposerons. Merci, cher collègue. à la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Olivier Cadic pour le groupe Union centriste pour six minutes. Monsieur

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, Monsieur le Ministre, bienvenue parmi nous et en tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, puisque ces français font partie de votre vos attributions, je vous dis combien nous sommes heureux et vous pouvez être sûrs que nous serons à vos côtés pour le bon accomplissement de votre mission. Nous examinons aujourd'hui le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'État du Qatar destinée à renforcer le cadre juridique de dos coopération militaire, le Qatar et la France entretiennent des relations bilatérales depuis la déclaration d'indépendance du pays en 1971, elles se sont développées au début des années 90 dans le domaine de la sécurité et des hydrocarbures, la volonté qatariennes de diversifier, pardon, l'économie du pays et de réduire sa dépendance à la rente gazière a permis d'élargir le spectre de nos coopérations à de nombreux secteurs dans le domaine économique, avec par exemple le métro de Doha que j'ai eu le privilège de visiter ouvrage exceptionnel issu d'un partenariat entre RATP Dev SNCF et un partenaire local, ou encore dans le domaine de l'aéronautique avec les Airbus, mais aussi dans les secteurs de la culture, comme le Musée national du Qatar conçu en forme de rose des sables par l'architecte Jean Nouvel encore dans le domaine de l'éducation, citons le lycée franco-qatarien Voltaire ou le lycée Bonaparte. Plus précisément dans le domaine industriel et de la défense, le Qatar et le 3ème, client de la France pour la période 2016, 2020, il représentait 18 % des commandes d'armes françaises en parallèle de ces contrats, des actions de formations sont dispensées aux forces armées qatarienne environ 230 qatariens ont été formés sur la base de Mont-de-Marsan et une quarantaine de soldats ont par ailleurs suivi des études dans les écoles militaires françaises, l'accord qui nous est présenté aujourd'hui, a été signé le 25 novembre 2019 dans le cadre d'une visite de Madame Florence Parly, alors ministre des armées, à Doha, il a été à adopté en commission le 9 janvier, il a pour but, donc de renforcer ce cadre juridique de la relation bilatérale de défense entre la France et le Qatar et ses dispositions s'appliqueront au personnel militaire ainsi qu'aux personnels civils, appelés à se déplacer dans le cadre de contrats d'armement. La coopération de sécurité de défense entre la France et le Qatar constitue un pilier de la relation bilatérale la signature le 4 mai 2015 du contrat portant sur l'achat de 24 avions Rafale, puis le déblocage de l'option pour 12 Rafale supplémentaires en décembre 2017 en sont l'illustration. Cela s'ajoute à l'accord destiné à accompagner les forces de sécurité qatariennes dans la préparation et la conduite de la Coupe du monde de football 2022, ce texte, qui nous avait été soumis par le gouvernement, a été adoptée le 15 février dernier par le Sénat. L'accord qui nous est donc présentée aujourd'hui renforce quatre juridique de nos coopération militaire avec le Qatar, l'absence de cadre constitue un réel frein à l'approfondissement de nos relations bilatérales, comme par exemple l'impossibilité de mettre en oeuvre, plus de la moitié des actions prévues par le plan annuel de coopération franco-qatarien, l'accord est équilibré, il est conforme à nos exigences constitutionnelles et conventionnelles. Cette précision est importante car cela a été dit. monsieur le ministre et je pense tous les sénateurs, la peine de mort. Et toujours en vigueur au Qatar. Car même si le pays applique depuis 2003 un moratoire sur les exécutions l'exécution d'un ressortissant népalais, condamné à mort pour meurtre en 2020 démontre qu'elle peut toujours être appliqué l'article 11 de l'accord protège les membres du personnel et les personnes à charge des 2 États contre la peine de mort et compte les traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Président du groupe d'amitié France-Pays du Golfe, j'ai eu le privilège de faire partie de la délégation qui a accompagné Emmanuel Macron pour ses visites de travail aux Émirats arabes unis dans l'État du Qatar et au Royaume d'Arabie Saoudite en décembre dernier. J'ai pu mesurer à plusieurs reprises la qualité et la profondeur des relations construite par le président de la République, entre la France et les monarchies du vol. Cela permet de concrétiser des résultats économiques spectaculaires qui renforceront l'emploi en France, le Qatar est un allié stratégique de la France dans une région connaissant de fortes tensions, un allié de la France dans la lutte contre le terrorisme, un allié au Sahel ou le Qatar a été d'un grand soutien logistique, un allié encore lors de l'opération Apagan en Afghanistan en août dernier. Comme l'a fait, la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées du Sénat, le groupe Union centriste votera donc pour ce projet de loi, je vous remercie.

Oui merci beaucoup monsieur le président, je voudrais simplement remercier les différents groupes pour leurs expressions et apporter peut-être juste à un élément de clarification à l'égard du président Gontard du président Laurent et du sénateur évidemment le Qatar est un partenaire stratégique de la France, mais le fait qu'il soit un partenaire stratégique de la France n'exclut pas que nous ayons sur certaines questions avec le Qatar, un dialogue continu et nourrie notamment sur les questions des droits humains en coopération avec nos partenaires européens dans le cadre des organisations internationales et c'est vrai également dans le cas de du droit du travail ou un certain nombre de réformes ont été conduites, notamment avec le soutien de l'OIT a d'ailleurs, ça a été mentionné à la tribune avec un certain nombre d'avancées, je pense notamment au salaire minimum et puis bien entendu, il y a encore certains nombres de progrès à accomplir, et le gouvernement sera évidemment très attentif à ce que dans le cadre de ce dialogue continu, constant et et nourri, hé bien ces progrès puissent continuer, il y a à se réaliser, il y a, dans le cadre des relations que nous entretenons avec l'État du Qatar merci. Merci, monsieur le Ministre, je vais mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, le vote sur article vaudra vote sur l'ensemble du projet de loi il y a-t-il des demandes d'explications de vote Madame Goulet. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame la rapporteure, mes chers collègues, moi je voterai pas cette convention, je la voterai pas ça changera pas grand chose au résultat on Marie a créé le groupe d'amitié avec les pays du Golfe, j'ai moi-même présidé ici il y a dans cette convention, monsieur le ministre, une avancée qui est importante par rapport au rapport que j'avais au

mais quand même, avoir tout ce soutien logistique pour un pays qui soutient pas seulement les talibans, mais aussi les frères musulmans alors qu'on travaille contre l'Islam politique me semble une hérésie complète, ne jamais avoir la moindre réserve sur les conventions signées avec le Qatar, y compris les conventions fiscales qui font de notre pays, un paradis fiscal pour le Qatar, me semble tout à fait inacceptable dans la période que nous traversons, je comprends très bien de Business as du jour, je comprends très bien le fait de vendre des armes, je pense que dans cette situation, on devrait être plus exigeant et je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue, il n'y a pas d'autres demandes d'explications de vote. Donc je mais aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'État du Qatar relatif au statut de leurs forces. Qui est pour. Qui est pour. Qui s'abstient. Le projet de loi est adopté définitivement. Chers collègues, je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour, la séance est suspendue.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2021. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire sur ce texte ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Gabriel Attal Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les sénateurs. Nous nous retrouvons pour l'examen du projet de loi de règlement et d'approbation des comptes pour 2021 après son adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, il s'agit d'une forme de passage obligé de la procédure budgétaire, ce texte ne fait ni plus ni moins que de prendre acte de ce qui s'est passé sur le plan budgétaire l'an dernier, mais c'est toujours un moment intéressant, d'abord pour mesurer le chemin parcouru et pour mesurer la dynamique et le chemin qui nous reste à parcourir, s'agissant de nos comptes publics 2021 a été au plan mondial, une année de montagnes russes sur le plan sanitaire avec des conséquences en chaîne sur la production, l'approvisionnement, et donc sur les prix, dans cet environnement marqué à la fois par la reprise et l'instabilité, l'exécution budgétaire de l'année 2021 illustrent les 3 principes qui, hier comme aujourd'hui, sont la boussole de infraction protéger relancée et maîtriser la reprise de l'économie française 6 8 % l'an dernier s'est établi un virgule 4 points au dessus de la moyenne européenne, ce dont nous devons collectivement nous féliciter, mai 2021 n'a pas été uniquement l'année du rebond plusieurs dérèglements sont apparues au fil des mois, certains sont liés aux résurgences épidémiques notamment la vague Omicron à l'Automne dernier et d'autres à la reprise, elles-mêmes en raison d'un phénomène de surchauffe économique, des règlements ont eu une conséquence nous faire redécouvrir le fléau de l'inflation que nous combattons vigoureusement pour protéger les Français, les tensions inflationnistes ne date pas de l'invasion de l'Ukraine, mais de l'Automne 2021 face à cette nouvelle donne, le gouvernement a réagi sans tarder, blocage des prix du gaz et de l'électricité indemnité inflation de 100 euros versés à 38 millions de personnes chèque énergie exceptionnel, ces mesures prises pour certaines dès septembre ou octobre 2021 nous ont permis de contenir les hausses qui pèsent sur le portefeuille des Français, même si nous savons que la situation est très difficile pour nombre d'entre eux, certaines de ces mesures ont bien sûr eu un impact Direct sur les finances publiques de l'année 2021, c'est la raison pour laquelle une seconde loi de finances rectificative, vous vous en souvenez a été présenté en novembre dernier, celle-ci prévoyait notamment l'ouverture de 3 8 milliards d'euros de crédits de paiement pour financer l'indemnité inflation que je viens d'évoquer ou encore celle des 600 millions d'euros pour le chèque énergie exceptionnel versé à 5 8 millions de ménages modestes en décembre dernier. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, un aperçu de l'environnement dans lequel nous avons évolué et des menaces que nous avons eu à affronter, mais tout au long de 2021, je le disais, 3 principes ont guidé notre action protéger relancée et maîtrisée protéger d'abord oui en 2021 nous avons poursuivi l'effort pour contrer les effets de la crise du Covid en adaptant constamment nos dispositifs au contexte sanitaire, économique, nous l'avons notamment fait au travers de de loi de finances rectificative adoptée en juillet et novembre qui ont ouvert près de 11,5 milliards d'euros de crédits supplémentaires, permettez-moi de partager avec vous, un constat les mesures de protection sanitaire assorties de restrictions d'activité décidée pour limiter la circulation du virus aura eu des effets plus dramatiques encore si nous ne les avions pas contré par de puissants mécanismes de soutien, je pense notamment aux fonds de solidarité et à l'activité partielle, que nous avons su mettre à disposition des acteurs économiques au bon moment pour ensuite les faire progressivement disparaître à mesure que la vaccination et le Pass sanitaire nous ont permis de lever les restrictions je pense également aux mesures qui nous ont permis de protéger le mieux possible le pouvoir d'achat des Français comme le financement de l'indemnité, inflation de 100 euros que j'évoquais il y a un instant ou la prolongation pour les étudiants boursiers du ticket eu à un euro, instauré depuis la rentrée 2020 sur le budget de l'État, ce sont 34 4 milliards d'euros de crédits qui ont été mobilisés l'année dernière sur la mission plan d'urgence face à la crise sanitaire composé de 4 programmes, celle-ci a notamment pu financer l'activité partielle, le fonds de solidarité pour les entreprises, le renforcement des participations de l'État au capital d'entreprises publiques, fragilisés par la crise, la compensation à la sécurité sociale des allégements de prélèvements pour les entreprises les plus touchés par la crise sanitaire évidemment l'achat de matériel sanitaire pour faire face à la pandémie, permettez-moi de partager quelques chiffres pour illustrer la manière dont nos dispositifs ont évolué au gré du contexte sanitaire et de la situation économique s'agissant de l'activité partielle le retour progressif au dispositif de droit commun s'était traduit par une baisse significative du nombre d'entreprises ayant bénéficié du dispositif au cours de l'année 2021 près de 500000 entreprises y ont eu recours contre un peu plus d'un 1000000 lors du premier confinement, ce qui est évidemment une bonne nouvelle puisque cela traduit une meilleure situation pour beaucoup d'entreprises en 2021 concernant le fonds de solidarité ce mécanisme traduit l'effort sans précédent conduit en 2021 pour répondre aux besoins des entreprises touchées par la crise sanitaire et mettre en oeuvre des aides plus ciblées, offrant une compensation pour les plus grandes entreprises, celles dont les coûts fixes sont particulièrement importants ou encore celle soumise à une forte saisonnalité, je pense notamment aux acteurs de la montagne pour lesquels un plan spécifique a été mis en place, ce sont ainsi près de 27 milliards d'euros qui ont été exécutés sur le programme en 2021, dit, des prêts garantis aux entreprises les femmes PGE ceux-ci recouvrait un engagement de l'État à hauteur de 93 milliards d'euros au 31 décembre dernier, soit une légère baisse par rapport à fin 2020, c'était alors 100 milliards d'euros, cette diminution est liée d'une part aux remboursements intervenus et, d'autre part à la diminution du montant de la provision pour risques d'appel en garantie, compte tenu de la nette amélioration de la situation financière des entreprises bénéficiaires, c'était tout l'objet de ces prêts garantis par l'État, protéger d'abord donc relancer ensuite, car l'année 2021, a été placée sous le signe de la relance et l'exécution budgétaire que nous vous soumettons en attestent, dans la période que nous avons vécu, l'enjeu n'était pas uniquement de parer à l'urgence, il s'agissait de préparer l'avenir, c'est ce que nous avons fait état protecteur donc, mais aussi État, stratège avec les 100 milliards d'euros du plan de relance mis en oeuvre depuis l'été 2020, je veux souligner devant vous là, scellé la célérité dans sa mise en oeuvre et les résultats obtenus, oui, nous avons su aller vite avec l'atteinte dès la fin 2021 d'un niveau d'engagement et de décaissements supérieur aux cibles qui avait été fixé, je le rappelle, fin 2021 72 milliards d'euros d'engagements 42 milliards d'euros de décaissement concernant ce plan de relance, je veux rappeler qu'un amendement a été introduit à l'Assemblée nationale en première lecture de ce texte à l'initiative du groupe socialiste, celui-ci prévoit la remise d'un rapport au Parlement en mai prochain, afin de permettre à la représentation nationale d'opérer un suivi sur le coût complet de chaque action et sous-action des 3 programmes de la mission, plan de relance, ouvert en 2020, 2021 et 2022 mais sans attendre mai prochain je veux d'ores et déjà partager avec vous un certain nombre de réalisations en matière de transition énergétique d'abord sur l'ensemble de l'année 2021 765000 ménages ont formulé une demande au titre de ma prime rénovent pour améliorer l'efficacité énergétique de leur logement, en matière de compétitivité ensuite en 2021 environ un tiers des entreprises industrielles françaises ont été soutenus, notamment à travers les dispositifs industrie du futur, près de 7900 entreprises bénéficiaires à fin 2021 dont et je veux le souligner 90 pour 100 de PME et de TPE ou encore le programme territoires d'industrie, plus de 1300 projets lauréats à fin 2021, je sais que vous envoyez dans chacun de vos départements, en l'occurrence, quand je me déplace sur le terrain, je rencontre à chaque fois des entreprises, des collectivités locales qui salue l'arrivée de ces dispositifs sur leur territoire en matière de cohésion, enfin, je veux souligner que l'année dernière 4 millions de jeunes ont directement bénéficié du plan, un jeune une solution, notamment grâce à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis qui a permis un flux d'entrée historique en apprentissage à hauteur de plus de 732000 jeunes à fin 2021, je veux rappeler qu'ils étaient moins de 300000 au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, en 2017, sans aucun doute, ces politiques ont puissamment contribué à la reprise de l'activité l'année dernière, permettant à la France d'être le seul grand pays européen à avoir retrouvé son PIB d'avant crise dès le 3ème trimestre 2021 certains évoqueront sans doute un simple effet de rattrapage après la contraction exceptionnel de notre PIB constatée en 2020, personne ne nie cet effet de rattrapage, mais admettons ensemble que son ampleur et que sa rapidité tiennent largement aux mesures de protection que nous avons mises en oeuvre maîtrisée enfant car des comptes bien tenus sont la condition sine qua non d'objectifs qui vont bien au delà des raisonnements financiers et qui garantissent notre indépendance, notre souveraineté et notre capacité à agir après un déficit public de 8 9 % en 2020, celui-ci s'est établi à 6 4 % en 2021, cette amélioration résulte largement du rebond de l'activité économique, que l'Insee a révisé à fin mai à 6 8 mais je veux l'encore souligné que le quoi qu'il en coûte, qui s'est imposé aussi longtemps que la situation économique, les l'exigeait, a joué un rôle décisif. Parce qu'il savait que l'État se tenait à leurs côtés, les ménages ont consommé et les entreprises ont sauvegarder l'emploi et ont investi. 1er point, cette croissance a été forte, parce que les acteurs économiques ont compris que la puissance publique jouer pleinement son rôle d'amortisseur 2ème point à la très bonne dynamique du marché du travail tient bien sûr à la croissance mais aussi aux réformes structurelles que nous avons conduite en matière d'assurance chômage, de formation professionnelle ou de renforcement de la compétitivité de nos entreprises, si bien qu'au 4ème trimestre 2021, le taux de chômage a atteint 7 virgule 4 % son plus bas niveau depuis 2008 2021 doit donc apparaître comme la première étape post-Covid sur le chemin qui doit nous conduire à ramener le déficit public sous la barre des 3 % en 2027, cet objectif est atteignable, je veux rappeler que nous l'avons atteint au début du précédent quinquennat pour la première fois depuis des années, cette dynamique vertueuse a été enclenché l'année dernière avec un reflux du déficit et des recettes fiscales plus élevées que prévu cette dynamique de maîtrise des comptes nous entendons la poursuivre durant ce quinquennat tout en maintenant les protections indispensables pour les Français les plus affectés par la hausse des prix notamment, je le disais, l'année 2021 a été celle d'un reflux du déficit public, passer de 8,9 % à 6 4 % malgré cette amélioration significative largement porté par le rebond de l'activité, le solde public reste dégradé en raison des mesures de soutien et d'investissements que je viens de rappeler devant vous, s'agissant du solde budgétaire, celui-ci s'établit à moins 170 7 milliards d'euros en 2021 en légère, je dirais : amélioration de 2 5 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2021 cela résulte notamment d'une hausse des recettes de 37,9 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2021 cette nette augmentation s'explique principalement par la reprise de l'activité économique en fin de 1er semestre, celle-ci se manifeste par des recettes supplémentaires perçus sur l'impôt sur les sociétés, plus 15,3 milliards d'euros sur la TVA, plus 10 milliards d'euros et sur l'impôt sur le revenu, plus 5 4 milliards d'euros, mais je vous le dis cela tellement le quinquennat qui s'ouvrent, ne sera pas celui du laisser-aller budgétaire Autrement dit, nous sommes passés de l'ère du quoi qu'il en coûte à l'air du combien ça coûte, comme l'a annoncé le président de la République, notre objectif est de ramener le déficit public sous les 3 % en 2000 s'agissant de la dette des administrations publiques, celle-ci a été ramenée à 112,5 % du PIB en 2021, après avoir atteint son plus haut niveau historique en 2020, c'était 114 6 % notre objectif est de la stabiliser en 2026 pour ensuite la réduire de façon graduelle, pourquoi faut-il ramener le déficit public en deçà des 3 % de notre richesse nationale et stabiliser la dette, non pas parce que ce chiffre serait un totem, non pas pour nous soumettre à je ne sais quel diktats d'abord parce qu'une grande nation honore ses engagements, nous avons des engagements à l'égard de nos partenaires européens et c'est une partie de notre crédibilité qui est en jeu, ensuite parce que sur le plan monétaire, nous sommes en train de changer d'époque, pour parler clair, ce qui est soutenable dans un environnement à taux d'intérêt faibles ne l'est plus quand ceux-ci remontent comme c'est le cas aujourd'hui, enfin, je veux rappeler que laisser filer les comptes, c'est se priver des moyens pour agir en temps de crise, et c'est justement parce qu'on a retrouvé des marges finale financière et des marges de manoeuvre financières grâce au sérieux budgétaire entre 2017 et 2020, que nous avons pu financer le quoi qu'il en coûte est-ce à dire pour autant que nous allons augmenter les impôts des Français non, nous les avons baissé de 50 milliards d'euros dans le précédent quinquennat et nous continuerons à les baisser, qu'il s'agisse des ménages, c'est une mesure du projet de loi de finances rectificative qui vous sera soumis dans les prochaines semaines avec la suppression de la redevance audiovisuelle, nous allons continuer aussi pour les entreprises avec la suppression de la CVAE pour continuer à baisser les impôts de production est dire que nous allons démanteler les mécanismes de protection alors que l'inflation fait rage non, nous allons les maintenir et nous allons même les renforcer pour et ceux qui en ont le plus besoin, avec les 20 milliards d'euros de mesures contenues dans le paquet, le pouvoir d'achat, examiné en ce moment même à l'Assemblée nationale et dont vous serez saisis là aussi dans les prochaines semaines, compris oui les prochains jours, vous l'aurez compris notre stratégie est claire tenir les comptes pour continuer à protéger les Français, tenir les comptes pour pouvoir financer les dépenses prévues imprévu et même imprévisible en tant que ministre des Comptes publics, je serai le gars le garant scrupuleux de cet équilibre et je sais que je vous trouverai à mes côtés, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. La parole est à Jean-François Husson rapporteur. Général de la commission des finances pour dix minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour la première fois depuis 22 ans, le gouvernement a déposé le projet de loi de règlement après le 1er juillet. Soit avec plus d'un mois de retard sur la date limite prévue par la loi organique relative au projet de loi de finances. Ce n'est pas un bon début pour vous, Monsieur le Ministre. Ce n'est pas un bon signal, voilà qui paraît en tout cas contradictoires au moment où le gouvernement dit vouloir travailler étroitement avec le Parlement, et alors que la révision de la loi organique a été l'occasion de rappeler l'importance de l'analyse de l'exécution budgétaire passer pour justement définir les orientations futures. Il a notamment été souligné ce matin en commission que les rapporteurs spéciaux n'ont pu travailler dans de bonnes conditions cette année. S'agissant du texte qui nous a été transmis, il convient de se réjouir que la France a effectivement connu un fort rebond de son activité économique en 2021. Il apparaît toutefois que le niveau global de l'activité n'est pas revenu en 2021 à celui qui était le sien en 2019, notamment à cause de la dégradation de notre commerce extérieur et d'une consommation encore déprimer. Par ailleurs, nos performances ont été moins élevées que celles de nos partenaires européens, nous appartenons en effet au groupe des quelques pays ayant connu un niveau d'activité inférieur à celui-là, dit 2019 pour les années 2020 et 2021. Ce rattrapage économique a eu un coup par ailleurs celui de la dégradation des comptes publics, monsieur le Ministre, en effet, si l'économie dans son ensemble a enregistré un montant de pertes de revenus cumulé de plus de 60 milliards, cela n'a été permis qu'avec l'absorption par les administrations publiques de 156 milliards d'euros de ses pairs. on peut observer que du point de vue économique l'année 2021 a finalement préfiguré un certain nombre de choc quatre que nous subissons en 2022 choc d'approvisionnement en matières premières choc sur l'évolution des prix choc sur les marges des entreprises et. Ce qui n'est pas le moindre choc sur le coût de financement de la dette, les prix à la production ont fortement accéléré au cours de l'année 2021, dans le contexte d'une reprise économique mondiale marquée. Les consommateurs n'ont pas immédiatement subissent cette augmentation, les entreprises ayant d'abord réduit leurs marges mais à compter de l'été 2021, l'inflation des prix à la consommation a fortement progressé et tout au long de l'année 2021, nous avons assisté à une remontée des taux d'intérêt nominaux des obligations souveraines à 10 ans qui sont passés par 2 fois en terrain positif. Les conditions de financement de la dette française change et il va, il va falloir en tenir compte pour l'avenir, dans ce contexte, la situation de nos finances publiques est la suivante : tout d'abord les recettes publiques ont été sous-évalués lors de l'examen du PLFR de fin de gestion en 2021 car, comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire, la prévision de croissance du gouvernement pour 2021 soit 6 25 % excessivement prudente quand en effet l'qui croissance était à lui seul égal à l'époque à 6 6 dans ce contexte, le gouvernement constate maintenant que les prélèvements obligatoires conduisent à un surplus de 30 milliards d'euros de recettes en réalité une prévision plus juste aurait divisé par 2 cette manne que le gouvernement brandit aujourd'hui comme un satisfecit de qualité de gestion. Avec 1460 milliards d'euros en 2021, les dépenses publiques sont inférieurs de 10 milliards à la prévision retenue au PLFR de fin de gestion toutefois ce montant nous éloigne très fortement des objectifs inscrits en loi de programmation des finances publiques. Ah si, mes chers collègues, en excluant les dépenses liées à la crise sanitaire et à la relance, soit environ 91 milliards en 2021, les dépenses publiques s'établissent à 55,4 % du PIB, contre 52,5 % attendu trois points de différence, le seul public s'établit à moins 160 7 milliards d'euros, soit 6,4 du PIB, il est d'ailleurs principalement supportée par l'État, tandis que les collectivités locales parviennent quasiment à l'équilibre et que les administrations de Sécurité sociale ont divisé par plus de 2 leur déficit. Notre endettement public diminue lui également d'environ 2 points de PIB mais reste à un niveau très important en comparaison européenne, je cite 112 9 % du PIB, soit, excusez du peu, plus de 40 points de plus que l'endettement de l'Allemagne éloquent. En outre, l'année 2021 et la première depuis longtemps où l'on assiste à une augmentation du poids de la charge de la dette, et cette tendance se poursuivra en 2022 puisque le PLFR pour 2022 que nous devrions examiner la semaine prochaine, prévoit une hausse de 17,8 milliards d'euros de la charge de la dette par rapport à la loi de finances, j'en reviens à présent au budget de l'État, dont le déficit s'établit en 2021 à plus de 170 milliards d'euros, c'est presque autant qu'en 2020, autrement dit un niveau historiquement élevé qui résulte à un niveau toute hausse historique des dépenses. Près de 420 milliards d'euros sur le budget général pour moins de 250 milliards de recettes. En fait, les recettes fiscales de l'État efface la forte chute, connu en 2020 et retrouvent leur niveau de 2017 alors même qu'une fraction croissante de TVA est affecté aux administrations de Sécurité sociale et aux collectivités territoriales la TVA était naguère une ressource majeure par dominante de l'État et ne lui rapporte aujourd'hui guère plus que l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les sociétés qui devait diminuer, selon la loi de finances initiale et finalement en hausse de 10 milliards d'euros par rapport à 2020, c'est d'ailleurs un exemple caractéristique des difficultés parfois de prévisions rencontrés par l'administration 2021. S'agissant des dépenses, elles ont augmenté de 37 milliards d'euros en 2021 et de 90 7 milliards d'euros en 2 ans c'est hausse résulte en particulier en 2021 du lancement de la mission 32 plan de relance, mais un grand nombre de missions du budget général sont concernés. Même si elle diminue la mission plan d'urgence face à la crise sanitaire consomme tout de même en 2021 plus de 34 milliards d'euros. Au total, et pour bien fixer les choses, le surcroît de dépenses entre 2000 19 et 2021 et plus de 3 fois supérieur aux sommes mises en oeuvre lors de la crise financière de 2008 à 2010. Or, je crains que le gouvernement ne considère le niveau actuel de dépenses comme un plancher pour les dépenses futures et non pas comme une situation exceptionnelle et temporaire puisqu'il n'a malheureusement fait aucune annonce jusqu'à présent, permettant de prévoir une diminution de certains postes de dépenses dans les années à venir, j'ai même entendu que pour ça, il comptait sur ces oppositions. Les dépenses de personnel du budget général de l'État, il use d'ailleurs, l'absence de mesures d'économies. Elles ont poursuivi leur augmentation tout au long du dernier quinquennat et les diminutions d'emplois prévue et promise n'ont jamais été réalisé. Si le nombre des emplois diminuent de près quatre 1000 et qui va longtemps plein travailler en 2021, c'est seulement en raison de difficultés de recrutement au ministère de l'Éducation nationale. Enfin, je déplore le montant assez extraordinaire des reports de crédits en 2021, monsieur le Ministre, plus de 36 milliards d'euros de report, alors que depuis l'entrée en vigueur de la LOLF le montant des crédits reportés chaque année avait toujours été inférieur à 3 8 milliards d'euros, le rapport est donc de un à 10, or cette pratique, qui devait être exceptionnelle car elle contourne l'autorisation annuelle des dépenses a été adopté comme norme par le précédent gouvernement, la quasi-totalité des crédits non consommés en 2021 ont été à nouveau reporté vers 2022 alors qu'il devrait être annulé en loi de règlement, le gouvernement considère-t-il cette pratique comme un acte de saine gestion des finances publiques, hé bien, alors qu'il s'exonère de règles organique, principe de spécialité d'annualité tout en appelant à la rigueur des comptes. à vrai dire, tout cela n'est pas très sérieux Monsieur le Ministre, il me semble que le projet de loi de règlement donne une vision quelque peu idéalisé d'une situation où l'accumulation des déficits creuse la dette au moment même où l'inflation et les taux d'intérêt repartent à la hausse, sans aucune perspective favorable de mesures qui pourrait conduire à rétablissement des comptes, en conclusion, la commission des finances propose de ne pas adopter le présent projet de loi de règlement. Comme je viens de l'indiquer, du point de vue de la procédure budgétaire, nous regrettons les opérations de report massif en fin d'année 2020 et 2021 et sans nécessairement conservé la destination initialement prévu des crédits ouverts. Par ailleurs, je rappelle que le seul n'a pas souhaité voter la loi de finances initiale pour 2021 dont le présent texte même révisé traduit l'exécution, le Sénat, après avoir voté les mesures d'urgence indispensable par pendant la crise sanitaire avait notamment contesté le choix du gouvernement de ne pas tenir compte de la dérive des comptes publics, par ailleurs, nous avions déjà appelé à privilégier des mesures temporaires puissante et mieux ciblé pour favoriser la sortie de crise dans le cas du plan de relance, ce sont les mêmes critiques que nous avons formulées lors du second PLFR pour 2021, à propos de votre premier chèque à 4 milliards d'euros, la fameuse indemnité inflation aussi compte tenu de l'ensemble de ces éléments à la fois pour les mesures que le budget exécuté comporte et les manoeuvres procédurales employée par le gouvernement en cours d'année, ce texte ne nous satisfait pas, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Isabelle briquet pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour cinq minutes.

Monsieur le président, monsieur le ministre à monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, monsieur le Ministre, dans l'exposé général des motifs de la loi du projet de loi de règlement soumis à notre examen, il est indiqué, je cite depuis 2018, le gouvernement a posé les jalons essentiels pour donner un nouvel élan structurant à cet exercice démocratique en lien avec le printemps d'évaluation instaurée par l'Assemblée nationale dans une logique de responsabilisation sur les résultats budgétaires et comptables, ainsi que sur la performance, conformément à la dynamique vertueuse prévue par la LOLF formulation sympathique mais il faut bien le relevé aux circonstances et ce à plusieurs titres le cycle électoral ne sera en effet justifier la transmission tardive de ce texte au mépris du temps parlementaire retourner ce retard pris aurait-il pu être mise à profit pour améliorer la lisibilité de ce texte et ainsi renforcer l'information parlementaire et citoyenne, là non plus, la clarté n'est pas au rendez-vous, j'ai bien noté la la satisfaction affichée du gouvernement quant aux résultats obtenus, notamment la réduction du déficit public, il faut bien dire qu'après une année 2020 particulièrement délicate : la comparaison des indicateurs ne peut s'en trouver qu'améliorer ce texte d'approbation des comptes ne saurait être mis au seul crédit de l'action du gouvernement telle qu'on voudrait nous le laisser croire les mesures mises en oeuvre sont en effet loin d'avoir porté leurs fruits crédit France relance sur 72 milliards engagés seulement 42 ont été décaissés, soit à peine plus d'un tiers du budget initial de 100 milliards d'euros, alors que la capacité de l'État, engager les dépenses est un enjeu fort de lutte contre la crise, d'autre part, on ne peut que noter le manque de sérieux et de sincérité dans l'exécution des comptes si les reports de crédits de 2020, 2021 était historique se constaté fin 2021 dépasse tout de même les 22 milliards cette façon de faire, ne met pas seulement le mal l'annualité budgétaire, elle a des conséquences bien réelles sur nos concitoyens ainsi le report de l'activité partielle un impact Direct sur le porte-monnaie des particuliers, si la consommation des ménages a progressé cette hausse n'a pas profité à tout le monde, loin de là, parallèlement à cela, côté recettes, l'État enregistrer 38 milliards d'euros de recettes exceptionnelles, là aussi, la sincérité budgétaire interroge quant à leur estimation initiale, alors même que ses recettes aurait pu, aurait dû servir à renforcer les services publics à répondre efficacement à l'urgence sociale, le gouvernement a préféré porter son attention sur les plus riches, baisse de la taxe d'habitation pour les 20 % les plus aisés, réduction des impôts, de production et ces baisses d'impôts ont d'ailleurs permis aux entreprises du CAC 40 de verser des dividendes des dividendes record à leurs actionnaires en matière de loi de finances, le en même temps on trouve rapidement ses limites, il n'est pas possible de faire en même temps des cadeaux fiscaux aux plus aisés et en même temps, attendre que les plus démunis puissent vivre dignement le ruissellement ne fonctionne pas, la loi du marché ne réduit pas les inégalités, elle permet juste d'enrichir ceux qui ont déjà beaucoup, en revanche, les services publics de proximité et l'hôpital éducation qui ont été délaissés sont les véritables armes contre la pauvreté, contre la précarité et pour garantir une vie digne à toutes et tous la politique fiscale du gouvernement et par ailleurs dans une impasse si le solde conjoncturel s'est en effet améliorée, force est de constater que le solde structurel c'est lui dégrader l'État ne peut ainsi durablement jouer avec les réductions d'impôts et se priver de certaines recettes fiscales avec mes collègues du groupe socialiste du Sénat, nous ne cessons depuis maintenant plus de 5 années de proposer le rétablissement de mesure de justice fiscale comme l'ISF devant les urgences du quotidien et les défis du siècle nous devons permettre à chacun de vivre dignement en garantissant l'accès à des services publics de qualité tout en permettant la transition écologique, ce projet de loi de règlement pour 2021 démontre le manque de sérieux du gouvernement et l'échec d'une politique qui n'a conduit qu'à accroître les inégalités fracturer davantage la société enrichir ceux qui n'en n'ont nullement besoin et sans pour autant faire preuve défaite d'efficacité économique entre report sous-exécution et annulations de crédits cette loi de règlement frôle même la sincérité dans son rapport, la Cour des comptes s'est d'ailleurs montré sévère sur ce texte, dénonçant au passage le mépris affiché, une nouvelle fois du Parlement et la remise en cause de sa mission de contrôle budgétaire, vous l'aurez compris ce texte en principe plutôt technique Marc tout à la fois la méthode et l'entêtement idéologique du gouvernement, le groupe socialiste, écologiste et républicain, votera contre ce texte. Merci, cher collègue, dans la suite de la. Question : la parole est à monsieur Didier Rambaud pour le groupe RDPI pour six minutes. Merci. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'entendais ce matin en commission des finances certains de d'entre nous parler d'une normalisation de la situation en 2021 je tiens avant tout à rappeler que cet exercice est marquée par les débuts du plan de relance ainsi que par le maintien des aides d'urgence au cours de PLFR ce que s'il fait face à une situation exceptionnelle qui s'est maintenu en 2021 à la nécessaire relance de notre économie, que tous, sans exception, sur ces bancs, nous appelions de nos voeux, face enfin au retour de l'inflation, nous avons agi, je voudrais ici rappeler le contexte exceptionnel qui a poussé le gouvernement ou quoi qu'il en coûte, alors que notre économie était mise en pause, les Français étaient pris en tenaille par l'effondrement de l'activité économique qui aurait pu affecter durablement le pouvoir d'achat, la situation sociale de notre pays s'annonçait sombre alors oui, nous assumons d'avoir soutenu les entreprises et les ménages, oui, nous assumons de ne pas avoir laissé l'économie française sombrer et entraîner une misère sans précédent, aujourd'hui refaire le match, après coup, beaucoup d'entre vous soutenez en dépit de nos divergences politiques, l'idée d'un soutien fort face à l'inflation et d'une relance ambitieuse, bien évidemment, il est plus simple de refaire l'histoire, une fois celle-ci terminée, je reprends ainsi les mots du député François Jolivet pour vous demander à quoi aurait-il donc fallu renoncer au rôti aurait-il fallu renoncer au chômage partiel, dont ont bénéficié tant et tant de nos concitoyens, en 2021 je crois, plus de 13 millions de salariés aurait-il fallu renoncer au fonds de solidarité qui a soutenu plusieurs milliers de nos entreprises après la crise sanitaire, nous faisons désormais face à un retour de l'inflation notamment causé par la reprise économique, la guerre en Ukraine, il y est pour beaucoup mais ça n'en est pas le déclencheur initial, je vous rappelle que l'inflation a commencé en Automne dernier, agir, la majorité présidentielle n'a pas attendu la crise sanitaire pour l'affaire. La loi pacte de 2019 était déjà une avancée notable dans l'amélioration des performances de nos TPE et PME d'un autre côté, la loi sur l'avenir professionnel à réformer l'assurance-chômage, l'apprentissage et la formation professionnelle en permettant aux entreprises de dépasser les obstacles qui les empêcher de se développer, nous avons soutenu la production en améliorant le pouvoir d'achat des ménages, nous avons soutenu la consommation, c'est le credo que nous avons défendu avant la crise et que nous continuerons de défendre dans les années à venir, force est de constater qu'il s'agit là d'une méthode qui marche soutenir à la fois la production et la demande constitue une réponse à l'endettement de notre pays funeste pour les perspectives de développement des générations futures, car ce n'est pas méconnaître les difficultés présentes que de rappeler que notre action a permis de faire baisser le déficit de l'État en dessous des 3 % avant 2020 en 2021 l'activité que économique a connu un dynamisme tels que les recettes fiscales nettes étaient en hausse de 37,9 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale permettant au déficit public d'être réduit à 6 4 % du PIB, là où il était de 8,9 % en 2020, une méthode que nous avons suivi depuis 2017 et avant que la crise ne frappe durement toutes les économies mondiales, cette méthode qui permet de promettre à nos enfants un monde juste, cette méthode, c'est celle qui m'a poussé à m'engager autrement en 2017, trouver des solutions pour simplifier, simplifier la vie des Français sans être déraisonnable pour nos finances publiques, c'est pour atteindre cet objectif que je me suis engagé et que je suis ici, c'est cet objectif que nous voulons désormais replacé au centre de notre politique, comme le soutient le ministre-Gabriel Attal, nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte, nous voulons désormais retrouver nos objectifs initiaux de finances publiques, c'est-à-dire. Tenir nos comptes en ordre, nous ne pouvons désormais engager de nouvelles dépenses sans qu'elle ne soit financé, nous voulons retrouver un déficit public inférieur à 3 % d'ici 2027 afin d'honorer nos engagements européens mais aussi et surtout afin d'honorer nos engagements nationaux, parce que c'est en menant une politique crédible et Vial est viable, que nous répondrons aux attentes et aux besoins des Français pour redire ce déficit, nous continuerons la stratégie d'emplois et de croissance que nous avons menées jusqu'ici, elle est la meilleure solution pour permettre à la fois de tenir nos comptes et de soutenir le pouvoir d'achat des Français et la capacité d'investissement des entreprises, je vous rappelle que la réforme de l'impôt sur les sociétés que nous avons porté génère plus de recettes fiscales, avec des taux plus faibles pour les entreprises, le taux de chômage de notre pays est au plus bas depuis 2008, cela démontre ni plus dis-moi l'efficacité de cette stratégie, poursuivons la stabiliser nos finances publiques passe également par une modernisation de celle-ci, c'est tout le travail que nous allons encore menées dans la continuité de la proposition de loi portée par les députés Saint-Martin Martin première étape dans nos réformes de la gestion des finances publiques s'adapter pour faire face aux changements et aux défis qui se dressent devant nous, telle a été notre action, telle est notre volonté est elle sera toujours notre vocation ces réformes que nous portons, s'inscrivent dans un projet résolument européen, il ne s'agit pas en effet de faire cavalier seul, ou contre les autres, mais bien en partenariat avec l'Union européenne, dont la commission a relancé récemment le débat sur la réforme des règles budgétaires de l'Union, les années de crise que nous avons connu resteront l'exception et l'objectif est désormais, à compter du PLF pour 2023 d'entamer l'assainissement de nos comptes publics d'affronter le retour de l'inflation et de poursuivre les chantiers entamés par le président de la République, l'avenir de notre pays en dépend et bien sûr, mon groupe votera ce projet de loi de règlement du budget Merci, cher collègue, dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Emmanuel Capus pour le groupe, les indépendants pour cinq minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission, mes chers collègues. Le 1er texte budgétaire de ce nouveau quinquennat porte sur le dernier exercice du précédent quinquennat c'est un état des lieux, une photographie de nos comptes publics, il pose une base de travail pour les 5 prochaines années. Ce projet de loi de règlement pour 2021 est aussi l'occasion de revenir sur les mesures prises pour faire face à une crise sans précédent. C'est l'occasion d'en dresser un bilan objectif je sais les critiques qui ont été émises sur la présentation tardive du texte, cette présentation a au moins une vertu, c'est que nous disposions d'un recul suffisant, l'analyse de l'année 2021 n'en sera que plus précise et lucide à cet égard, 2 évidence s'impose : la première c'est que nos finances publiques ont été lourdement impactée par la crise sanitaire, la seconde tient à la situation dans laquelle nous avons abordé cette crise malgré les efforts du gouvernement pour maîtriser le les comptes au début du précédent quinquennat nous sommes toujours devancée par l'Allemagne qui a remis de l'ordre dans ses comptes dès 2012, nous avons du retard. Notre taux d'antenne d'endettement s'établit ainsi à 113 % du PIB fin 2021, soit une amélioration de 2 points par rapport à 2020 outre-Rhin, la dette publique est contenu sous la barre des 70 % du PIB et pourrait prochainement revenir dans les clous de Maastricht. Notre déficit public à 6,4 % du PIB reste alarmant, même s'il s'améliore nettement par rapport à 2020, cependant, la cote d'alerte est atteinte, pourtant de nombreux indicateurs nous autorisent à un optimisme raisonné la croissance avoisine les 7 % un score digne des 30 Glorieuses le chômage lui avoisine les 7 % un taux historique au plus bas depuis 2008, comme vous l'avez dit, monsieur le Ministre, mais même à l'exception de début 2008 depuis le début des années 80 avant les années Mitterrand. Ce dynamisme se ressent dans les recettes de l'État, elles ont augmenté de 37 milliards par rapport à la dernière loi de finances rectificative pour 2021, c'est une bonne nouvelle, nous aurions tort de faire trop de politique, mes chers collègues sur ce texte qui a qui avant tout une formalité comptable cependant nous aurions également tort de nous voir dans ces bons résultats, de ne pas voir dans les bons résultats, les effets de la politique menée par le gouvernement pendant la crise, les 34 milliards d'euros mobilisés en 2021 dans la mission plan d'urgence face à la crise sanitaire ont préservé l'économie, ils ont permis à la fois de sauvegarder les emplois et les entreprises, au plus fort de la crise et de renouer rapidement avec la croissance dès la levée des restrictions sanitaires mais c'est précisément ce Stop and Go, sanitaire, comme vous l'avez dit, à juste titre, Monsieur le Ministre, c'est ce Stop and Go mondialisée qui a causé dès 2021 l'inflation dont dont nous subissons aujourd'hui les pleins c'est fait la guerre en Ukraine a fait en réalité qu'aggraver la situation, le gouvernement avait d'ailleurs. Réagir rapidement dès les prémices de cette inflation avec le bouclier tarifaire pour contrer la hausse des prix de l'énergie et le chèque, inflation, notre groupe a soutenu ces mesures. Généralisé en 2021, elles ont pour ainsi dire clos l'ère du quoi qu'il en coûte, car l'inflation a désormais pour conséquence la hausse des taux d'intérêt emprunter aura de nouveau un coup nous ne pourront plus agir dans le futur, comme nous l'avons fait en 2021 il faudra cibler les dispositifs d'urgence sur les plus fragiles, mais j'anticipe déjà sur les prochains débats. Je relève simplement ce tournant qui me semble bienvenu, j'avais proposé avec mon groupe lors du dernier pff. C'est-à-dire de conditionner chèque inflation aux revenus du foyer, vous me direz, Monsieur le Ministre, qu'on a tort quand on a raison trop tôt mais ça au Sénat, nous le savons, nous ne En tout état de cause, mes chers collègues, c'est une page qui se tourne, avec ce projet de loi de règlement, celle du quoi qu'il en coûte, et nous le voterons donc en responsabilité et ce d'autant plus que comme vous l'avez rappelé : il ne s'agit que d'un dernier acte de la réalité de nos comptes publics. Il faudra en revanche bientôt engager le désendettement de l'État et nous y prendrons Monsieur le Ministre, toute notre part. Je vous remercie. Merci, cher collègue, dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Jérôme Bascher pour le groupe Les Républicains pour sept minutes. Monsieur

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, dit donc, vous n'avez pas de chance, Monsieur le Ministre on vous a caché la réalité des comptes dans la mandature d'avant, non sur la forme, sur le fond comme sur les fonds, vous n'êtes pas. Vraiment sur la forme, comment voulez-vous. Que les Français respectent la loi, lorsque le gouvernement ne respecte pas, excusez du peu, les lois organiques. Vous vous êtes dit le garant des comptes, je vous ai écouté, je vais vous répondre le garant des comptes mais pas le garant de la loi, en tout cas, hein, parce que vous ne respectez pas donc ça commence pas très bien mais il faut bien commencer. Est-il normal qu'un gouvernement, certes sans majorité absolue ne votent la loi de règlement pas dans les délais de rigueur. La loi de finances rectificative et le rapporteur général a souligné tout à l'heure. Pardon, De 36 milliards la Cour des comptes, vous avez demandé d'arrêter cela, hé bien hop en 2021, certes, c'est un petit peu moins c'est 27 milliards d'euros, excusez du peu, c'est 3 milliards huit là le plafond, mais on ne peut pas continuer comme cela, monsieur le ministre. La Cour des comptes, vous l'a dit une fois, vous refaites de fois, il y aurait un vrai magistrats financiers, le gouvernement serait déféré devant le le procureur financier. Car, par 2 fois vous violer expressément la loi organique sur les dates sur les plafonds. Vous vous êtes dit aussi que vous étiez le garant des engagements européens. Mais enfin, c'est le ministre, il arrive quand le programme de stabilité. Tous les pays européens ont transmis le programme de stabilité à Bruxelles, tous les pays européens et nous. On ne voit pas de fumée bleue, donc on attend la date, monsieur le ministre espère que vous nous répondrez alors là encore sur les comptes de concours financiers, vous ne respectez pas les règles des comptes de concours financiers, c'est aussi des règles de la loi organique, je sais bien, on viole tout ça à bras comme ça à bras raccourcis tout le temps, allez hop tout ça, ça passe inaperçu, on s'en moque, mais qu'est-ce que c'est que cette direction que vous avez, Monsieur le Ministre, pour mettre un peu d'ordre, ils ne savent plus, ils ont oublié la loi organique votée à l'unanimité, les 2 assemblées, on oublie, il serait peut-être le temps de respecter la loi, enfin, et je vous l'avez dit en commission des finances, le fait est, c'est la 2ème année consécutive que vous supprimiez des emplois dans les lois de règlement, ce n'est pas acceptable quand on supprime des emplois, on l'annonce on ne le fait pas, comme cela, ah bah oui.

regardez bien les la la loi de programmation des finances publiques, regardez bien le rapport du Haut Conseil des finances publiques, il montre bien que la divergence a lieu en 2019 elle diverge gravement et c'est pour cela que nous arrivons dans une telle circonstance alors sur les recettes, regardons bien ce dont il s'agit 195 milliards de recettes fiscales 285 milliards de dettes. émises 51 % de nos ressources par un impôt 49 % par la dette, voilà la réalité de ce qui est, aujourd'hui, j'avais dit, lors du vote, souvenez-vous ici. Exceptionnellement, j'avais pris la parole, alors qu'en principe pour la pompe sur ce vote là que on allait financer à 50 % par là d'être notre budget. Nous y sommes, enfin, vous nous avez dit. Protéger relancer maîtriser, c'est l'utilisation des fonds, alors je vais commencer par maîtriser, bon bah les gens, on ne maîtrise pas la charge de la dette, hein, ça, on a bien compris que ça c'était pas tellement le truc, hein, on était passé de 35 8 milliards à 37 virgule et sur l'effet volume sur l'effet volume, il y avait déjà la dette. Qui augmentaient l'augmentation qui sourde est derrière cela. Les appels en garantie, c'est très bien, chemise, vous les avez évoqués : moins 2 milliards 5 mais attendez les appels en garantie, on a décalé les PGE et demandé aujourd'hui à la Banque de France qui est en train de calculer un peu frénétiquement savoir où ils en sont, parce que c'est en 2023 avec l'effet d'inflation, les marges qui auront été supprimés, que les PGE devront être remboursés, et là on verra s'il y a pas de défaillances d'entreprises. Alors, faites bien attention, faites bien alors après, vous avez dit oui relancer bah oui d'accord, vous avez relancé pour 18 8 millions les dépenses supplémentaires en 2021 milliards pardon milliards excusez-moi, merci monsieur le président. Les dépenses pilotables elles, elles ont augmenté de 7,1 milliards et puis après, les autres dépenses de 18,6 milliards donc autant pour la relance que pour les autres dépenses, en fait, il n'y avait pas de relance, il n'y a pas de maîtrise. De la dépense publique, voilà la vérité, et donc il faut bien le dire, vous avez voulu dire qui vous maîtrisiez vous ne maîtrisez pas, y compris dans la relance et enfin protéger. Monsieur le Ministre pas protéger, protéger quoi, vous savez que nos armées aujourd'hui après que nous avons heureusement et l'Ukraine, en fournissant des armes. En fournissant des munitions. Bah, nous ne sommes plus. Et c'est bien ça le sujet, sommes-nous armée sans polémique, mais le Sénat l'avait dit, notre collègue Jean-Pierre Vogel, dans un rapport de 2019 du Sénat ou Bruno Belin tout à fait récemment dans sa commission, sommes-nous armé pour lutter contre les incendies, non, on l'avait dit, c'était la commission des finances en 2019, le rapport de Jean-Pierre Vogel. Hé bien, sommes-nous aussi armé pour l'hôpital, sommes protégeons-nous les Français de cette façon-là, protégeons-nous les Français de l'insécurité réelle, non la loi pour le ministère de l'Intérieur, elle est toujours pas voté monsieur le Ministre, non donc vous avez les affaires étrangères, j'avais oublié, il y a eu un excellent rapport fait part de, de nos collègues qui vient d'être rendu récemment sur le corps diplomatique et les problèmes que cela posait non tout sur tout le surtout sur l'hôpital sur la santé, vous n'avez pas protégé les Français, les résultats sont là, et donc c'est bien cela que je trouve dommage dans vos propos, alors j'en termine monsieur le Ministre. Certes, Certes, les élections vous auront reconduit, vous avez flatté et permettez que je fasse le même reproche à votre budget que celui que Spinoza faisait au régime monarchique, c'est pousser les Français à combattre pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut.

président. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission chers collègues. Le groupe écologiste solidarité et territoires votera contre ce projet de loi de règlement du budget et ceci pour 2 raisons principales. Tout d'abord, ce rapport constate un budget 2021 traduisant son inefficacité pour réduire les inégalités dans notre pays, disant cela, Monsieur le Ministre, nous ne nions pas la nécessité des bouclier tarifaire et d'autres mesures, venus en soutien, même tardif, aux ménages les plus modestes. Mais nous déplorons la logique de votre majorité de répartition des richesses qui globalement âge quelques chèques aux plus vulnérables et offrent des réformes fiscales, structurelles au bénéfice des plus aisés. Nous voterons contre ce rapport également car il révèle l'inefficacité de vos actions en terme de bifurcation écologique, j'y reviendrai. Il est entendu que nous sommes là pour constater des résultats financiers et que l'exercice pourrait se vouloir plus comptable que politique. Mais les chiffres que nous sommes censés approuver aujourd'hui témoigne bien des choix politiques de votre gestion libérale. Pourtant, Monsieur le Ministre, je vous l'accorde, la situation des entreprises nécessitait soutient en cette période de pandémie, en particulier pour les milliers de TPE, PME de notre pays fragilisé par les crises successives. Mais les entreprises du CAC 40 ont distribué en 2021 57 1 milliards de dividendes, c'est un record absolu en hausse de 33 %, c'est du jamais vu, avait-elle besoin dès lors de recevoir des aides publiques, elles qui ont par ailleurs supprimer 27613 emplois cette même année 2021 et dont les patrons ont par ailleurs augmenté de 23 pour % le rémunération les portant à 237 millions ça ne vous choque pas, hé bien nous, ça nous choque terriblement l'argent public versés à ces grands groupes, n'a pas nourri l'emploi, il a enrichi les actionnaires. Les conséquences de ce budget sont un accroissement des inégalités entre ceux qui accumulent richesse des profits et ce dont le travail est notoirement sous-payés qui peine à se nourrir à se loger à offrir des vacances à leurs enfants à vivre tout simplement dignement rendez--vous social manqué donc et rendez- vous manqué également avec l'indispensable bifurcation écologique. Monsieur le Ministre, première question : pourquoi avoir supprimé 2062 équivalents temps plein des effectifs du ministère en charge de l'environnement en 2021, si c'est une priorité. 2ème question quand près de 12 millions de Français sont concernés par la précarité énergétique n'est-ce pas problématique que 4 5 milliards d'autorisations d'engagement du volet écologie du plan de relance n'aient pas été consommé. Quant au budget vers présenté comme une innovation majeure. Il évalue trop peu, trop mal et ferme les yeux sur certaines dépenses néfastes exonérations de taxation du kérosène ou bien les milliards d'euros, qui finance les entreprises des secteurs polluants, sans aucune contrepartie écologique ni sociale, comme le soulignait d'ailleurs récemment ATD quart Monde, le Secours catholique Caritas France et le réseau Action Climat dans ce budget Vert qui est un budget essentiellement de communication 93 % des dépenses de l'État, au sens large, ont un impact environnemental neutre ou non côtés qui peut y croire, il conviendrait plutôt Monsieur le Ministre, d'appliquer la loi 2015, sur les nouveaux indicateurs de richesse loi et là, ce qui n'est plus appliquée depuis 2018, comme le rappelait ma collègue députée Éva Sas, la semaine dernière au Palais Bourbon, il serait intéressant de savoir quelle a été l'impact des 488 milliards d'euros de dépenses publiques de 2021 sur l'espérance de vie en bonne santé, sur le taux de décrochage scolaire sur l'empreinte carbone de la France ou sur les inégalités de revenus. Pour conclure un mot sur la dette publique et le déficit budgétaire non, Monsieur le Ministre des Finances nous rappelle et vous le faites également Monsieur le Ministre, très fortement qu'ils ont atteint la cote d'alerte. Une autre cote d'alerte est atteinte, c'est celle de la dette climatique, les incendies se multiplient sans que malgré le dévouement de nos pompiers notre capacité d'y faire face est évolué comme le président Larché vient de le constater. Les inondations sont aussi puissantes à la Roya et ailleurs, que les sécheresses sont graves persistante et structurel dans plusieurs dizaines de départements les canicules se succèdent, mettant à mal les plus fragiles d'entre nous, mais aussi les productions agricoles et l'ensemble du vivant, animal et végétal, 100 des oiseaux et 67 % des insectes ont disparu et des milliers d'espèces sont menacées, selon Lipper BES 4 centrales nucléaires viennent d'obtenir une dérogation aux règles environnementales pour préserver leur production au détriment de la biodiversité, chers collègues, oui, la cote d'alerte est atteinte, mais pas seulement au plan financier, nous devons ensemble franchir le cap de la transition écologique, c'est une urgence vitale pour notre société, comme pour la planète. Chers. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Pascal Savoldelli pour le groupe CRCE pour cinq minutes. Merci monsieur le président, c'est le ministre mais Sharp, mes chers collègues alors passer du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte vous nous suggérez comme ministre du Budget. Et je vous le dis, Monsieur le Ministre, il faut peu de mots pour exprimer l'essentiel. Mais il faut tous les mots pour le rendre elle. L'heure est venue plutôt de passer du quoi qu'il en coûte pour les finances publiques, oh, qui doit payer. C'est ça l'esprit de responsabilité. Et l'opposition de gauche au gouvernement mais aussi à la majorité sénatoriale s'inscrit dans une double légitimité, celle tirée de l'élection et celle de la qualité de l'argumentation. Ce projet de loi de règlement et l'occasion de montrer que vos propositions sur le pouvoir d'achat insuffisante au demeurant, ne sont pas financés. Le président de la République avait brandi l'économie de guerre ses ministres entonnait le trésor de guerre, la communication était bien rodé, mais ça ne risque résiste pas à l'épreuve des faits par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale, le solde budgétaire de l'État n'est supérieur que de 2 6 milliards, difficile d'y voir un trésor de guerre, la vérité, c'est que les recettes fiscales ne font que revenir à leur niveau des années 2017 et 2018 encore là, difficile d'y voir un trésor de guerre et à seulement 2 mois de la fin de l'exercice comptable sans explication pour une bonne part d'entre elles, les recettes fiscales connaissent un écart de 18,2 milliards c'est toujours pas un trésor de guerre. S'agit-il, Monsieur le Ministre, d'un recours électoraliste à des mécanismes strictement comptable, la question vous est posée. La taxe sur les produits énergétiques, notamment sur les carburants a été dopé par la hausse des prix a désormais reversées au budget général sans que rien ne se passe les 6 8 milliards qui augmente les recettes fiscales, le dernier acompte d'impôt sur les sociétés, marque un rebond de 10 1 milliard, signe que l'activité serait florissante mais, là encore après une récession après la récession parmi les plus importantes d'Europe, et vous le savez bien, le dernier raconte dépend du versement des précédents estimé à partir de 2020, donc l'impôt des sociétés progressent en 2021, parce que l'activité en berne en 2020 à minorer les premiers versements donc pas de trésor de guerre du côté des dépenses, les sous-consommation alors la demeure à des sommets, 24 6 milliards d'euros, dont un tiers n'a rien à voir avec la crise sanitaire, ou encore le plan de relance, autrement dit, je le dis à l'ensemble des collègues 5,5 % des crédits que nous avons voté ici ne serve in fine et à rien si ce n'est d'améliorer artificiellement le solde budgétaire lorsqu'ils sont reportés ou annulés les principes budgétaires les principe d'annualité et de spécialités ont été passablement sapée par le quinquennat précédent Monsieur le Ministre, la situation exceptionnelle, n'en est pas la plus plus grande cause Monsieur le Ministre, je vous le redis on aura qu'avant de se revoir, mais la démocratie représentative et les finances publiques, ce n'est pas incompatible. Les exemples sont nombreux en recettes et en dépenses qui ne permettent d'affirmer que ceux qui veulent voir dans les résultats comptables dans les 2021 trésor de guerre sont insincère. Nous tenons à rassurer la majorité sénatoriale, alors je vous rassure : pour le capital, impossible de voir en le ministre Atal ou son collègue, le ministre Lemaire des belligérants le capital peut dormir tranquille et du quoi qu'il en coûte aux qui doit payer, vous disais-je, et pour cause les 50 milliards de baisses d'impôts de votre quinquennat dont 15 virgule 3 milliards pour la seule année 2021 vont se répercuter inexorablement sur les recettes fiscales de l'État, alimentant un déficit structurel j'ai bien dit un déficit structurel pas conjoncturel qui ne cesse de croître, il est temps de se poser, je sais ce que j'appellerais les questions qui dérangent, mais comment expliquer que l'excédent brut d'exploitation des entreprises 564 6 milliards en 2021 pour un impôt sur les sociétés, brut de 74 5 milliards soit amputée de moitié à cause des niches fiscales et dégrèvements en tous genres 2ème question qui peut éventuellement dérangé, comment expliquer que depuis le début du quinquennat près de 40 pour 100 du produit, TVA impôt injuste par excellence, ne sert plus à financer des services publics de l'État mais alimente vos exonération d'impôts et de cotisations en tout genre et puis aller 3ème question comment expliquer que les collectivités territoriales soient obligés de quémander à l'état des moyens financiers pour pouvoir administrer les services publics du quotidien et financer les investissements, par exemple dans les écoles, les stades, la voirie et bien d'autres réalisations enfin comment enfin expliquer que vous rappelez nous rabâcher les oreilles alors tantôt avec le désastre annoncé, tantôt vous nous parlez de la côte d'alerte pour évoquer quoi la dette publique. Mais la loi de finances après loi de finances sur les 3 dernières années, Monsieur le ministre. J'ai pu mettre en doute la sincérité budgétaire ou l'un plutôt l'insincérité budgétaire de votre gouvernement et là, il faut parler avec responsabilité et bien évidemment respect mais l'envolée de la dette publique, c'est votre responsabilité, vous présenter un projet sur le pouvoir d'achat qui constitue une base de discussion mais les manoeuvres du calendrier de présentation des comptes Dolan et pour les décalé après la séquence électorale n'y changeront rien à la dette publique financera les mesures de pouvoir d'achat aux Français, donc il est facile de comprendre dès lors les raisons pour laquelle le renouvellement des méthodes démocratiques au Parlement n'aura pas lieu le débat va être clos avant qu'il commence donc vous comprendrez bien évidemment que notre groupe, le groupe CRCE aura hein, non pas de droite, mes chers collègues, mais un non de gauche à votre projet de loi, merci de votre attention. La parole est à Vincent Capo Canellas pour le groupe Union centriste pour trois Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le marathon budgétaire de cette session extraordinaire débute avec ce texte de loi de règlement, il débute tardivement et on peut le regretter, même si les rapporteurs spéciaux de la commission des finances ont pu livrer leurs analyses, j'observe également que nous devrons attendre la rentrée pour connaître votre vision pluriannuelle, l'objectif des 3 % déficit en 2027 gagnerait sans doute être rapidement documenter, mais commençons d'abord par 2021 l'année 2021 a été con, c'est le moins qu'on puisse dire, ce projet de loi de règlement et d'abord le reflet d'une situation exceptionnelle. Situation qui a justifié des efforts budgétaires immédiats et importants, nous y sommes sensibles, on peut en effet lire les chiffres d'abord en positif, les recettes ont largement augmenté en 2021 plus 38,2 milliards avec une progression des recettes fiscales de 39 8 milliards la poursuite des baisses d'impôts. Taxe d'habitation, impôt sur les sociétés et la baisse des impôts de production décidées dans le cadre du plan de relance sont à noter comme élément favorable : les recettes fiscales ont connu une progression hors mesures nouvelles de 18 % nettement plus élevé que le PIB et donc on peut en déduire que les baisses d'impôts sont positives pour l'activité et les recettes, les recettes fiscales ont été supérieurs de 18, il a 2 milliards la prévision de la loi de finances rectificative, on peut sans doute s'en réjouir comme s'interroger sur la prévision néanmoins en négatif, les dépenses de l'État ont progressé très fortement du vingt-et-un et la raison ne tient pas uniquement aux mesures d'urgence et de relance, les dépenses ont augmenté de 90 milliards sur les 2 dernières années 53 virgule 6 milliards en 2020, 37 virgule 1 milliard en 2021, les dépenses du plan de relance 17 17,5 milliards pèse bien sûr, comme la mise en place de l'indemnité inflation 3,3 milliards comme le nouveau palier la loi de programmation vidant militaire, pardon, de 7 milliards et plus inquiétant, l'augmentation de la charge d'intérêts de la dette de milliards déjà l'année dernière en négatif encore la Cour des comptes, rejoint cette fois à la commission des finances vous constater plusieurs entorse aux règles budgétaires s'agissant de l'annualité des autorisations de programme, les autorisations de dépenses et la spécialité des crédits, les crédits reportés fin 2020 36 virgule 7 milliards et fin 2021 23 2 milliards sont importants. Des crédits votés sur des programmes budgétaires ont parfois être financer des dépenses d'autres programmes la portée des votes du Parlement est ainsi affaibli au total la sortie progressive de la crise du Covid, a justifié que le quoi qu'il en coûte affecte encore nos finances publiques sans doute fallait-il agir pour faire face aux crises, mais nous devons nous poser la question du financement de ses efforts, le ministre des Finances a parlé lui-même de cote d'alerte le 1er président de la Cour des comptes devant notre commission des finances la semaine dernière à lui lancé un message d'alerte, il y a de quoi l'augmentation significative de la dette, nous a conduit à la fin 2021 à plus de 2800 milliards d'euros, en hausse de 150 milliards par rapport à 2020 et de 430 milliards par rapport à 2019, des chiffres qui donnent le tournis, même si la France a connu une relance de l'activité économique de 6 à 8 % en volume, soit la plus forte depuis 1969 nous ne pourrons pas baser notre stratégie de maîtrise de la dette sur la croissance encore au moins au moment où celle-ci faiblit, le rapport de la Cour des comptes est à cet égard une alerte supplémentaire, ça veut dire aussi que pose la question de la souveraineté financière de notre pays, c'est ce diagnostic qui conduit la majorité du groupe Union centriste à s'abstenir sur cette loi de règlement d'autres votes pour l'essentiel favorable s'exprimeront et je pense que le président de elle aura l'occasion d'exprimer sa vision merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Christian Billac pour le groupe RDSE pour cinq minutes.

Monsieur le président. Monsieur le Ministre. Afghanistan. Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous réunis pour un exercice annuel obligé et combien il est important, le règlement du budget l'approbation des comptes de l'année 2021 une année caractérisée par une crise, déjouant toutes les prévisions et par le sceau de l'incertitude aujourd'hui la certitude semble devenue une certitude en matière d'orientation budgétaire, mais pas seulement, gouverner c'est prévoir, mais prévoir devient un exercice de plus en plus aléatoire, sans visibilité sur l'évolution à court terme et sans pouvoir en mesurer pleinement les conséquences. Pourtant, nous devons garder en tête l'objectif du redressement des finances publiques car je me permettrai de citer un nouveau mandat France les comptes désordre la marque des nations qui s'abandonnent. Le projet de loi et de règlements d'approbation des comptes pour 2021 et s'articule autour de 8 articles avec l'article liminaire, qui présente l'effort structurel conjoncturels affectif après l'exécution du budget com aux hypothèses de la loi des finances et de la loi de programmation.

le soir le c'est un bidon qu'à 4,4 % du PIB au lieu des 0 5 autorisé par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Le déficit budgétaire de l'État devient abyssal, avait 170,7 milliards d'euros améliorer de 34 milliards par rapport à la seconde loi rectificative. Le budget général est en déficit de 171 milliards et demi et les recettes sont en hausse de 27 vers de 3 milliards par rapport à la 2ème loi de finances rectificative. à ce sujet, il convient de noter que les finales, les recettes fiscales ont retrouvé leur niveau d'avant-crise, hein Rochatte honnête et au même progressé de près de 30 milliards par rapport à 2018. Recettes brutes mais cette bonne nouvelle n'améliore malheureusement pas notre situation financière. D'ailleurs l'article Dow démontre le besoin de financement de 285 vers virgule 7 milliards de déficit, financé par l'émission d'une autre date de 260 milliards d'euros à moyen et long terme. On continue avec l'article 3 qui présente un résultat de moins 142 milliards d'euros et un bilan un déficit, il y avait 4 milliards d'euros. L'article IV continue à faire apparaître des dépenses brutes, un autre stage le 4 milliards, 655 milliards d'euros les principales missions de dépenses en crédits de paiement par action comprise reste l'enseignement, la défense, les engagements financiers de l'État et le plan d'urgence sanitaire. Les articles 5 aussi sur l'exécution des Budgets annexes et des comptes spéciaux hors FMI sont en amélioration de sacs le 9 milliards toujours par rapport à la seconde loi de finances rectificative avec le solde de 0 8 contre au moins 5,4 en 2020, le compte d'opérations monétaires, le FMI est à découvert le dix-sept faire de 3 milliards d'euros. L'article 7 prévoit l'annulation de la dette de l'État somalien 24 millions d'euros, conformément à un accord bilatéral que nous avons signé en 2020. Chers collègues, si ce projet de loi, le règlement retrace une année 2021 marquée par la crise. On peut regretter que certaines dispositions n'aient pas été adopté afin de commencer à retrouver le chemin vers des finances saines, des collectivités territoriales, reste les grandes aux oubliés du fameux, quoi qu'il en coûte. Malgré leur rôle essentiel dans la gestion de la crise sanitaire et dans la reprise économique. Leur donnera tort en fait les moyens pour agir au plus près de nos concitoyens. Nous avons entendu le Sénat va majoritairement rejeté ce texte avec des mots, des sur des Selon les bancs en ce qui concerne les membres du groupe RDSE, ils vont se partager entre abstention garde option en attendant de connaître les attention du budget 2023 à la rentrée, et nous espérons, monsieur le ministre, que les critiques que j'ai pu émettre seront écoutés par votre gouvernement, je vous remercie. Merci, cher collègue, dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Rémi Féraud, pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour 4 minutes.

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, comme chaque année donc, le temps nous est compté, puisque nous y consacrons un temps très court à l'examen du projet de loi de règlement, la présentation du texte par le gouvernement accuse en plus un retard justifiée par des arguments qui, on l'a vue n'ont convaincu personne qui montre le peu de considération pour le temps parlementaire ce que nous regrettons, et comme l'a dit ma collègue Isabelle briquer les sénateurs socialistes vont donc voter contre ce projet de loi de règlement, il y a plusieurs raisons pour cela qui recoupent en partie mais en partie seulement celles exposées par le rapporteur général au nom de la commission des finances, d'abord sur la question de forme qui est quand même très révélatrice, ce texte nous arrive plus d'un mois après la date à laquelle la loi organique impose son dépôt, le nouveau gouvernement affirme vouloir favoriser le dialogue avec les parlementaires, cela ne pour l'instant qu'un simple voeu je pense que ce retard pose ou à poser un problème démocratique car dans les règles et dans les temps, ce texte aurait été aussi un objet intéressant pour le débat de la campagne législative, S. Monsieur le Ministre, ce que le gouvernement a voulu éviter et juste après avoir fait adopter en fin de quinquennat une loi organique de gestion des finances publiques qui visent à améliorer l'information et le contrôle du Parlement, vous conviendrez qu'il y a là une contradiction, ensuite, nous n'avons pas au groupe socialiste, l'habitude de voter chaque année contre la loi de règlement, mais comme l'année dernière l'exécution s'éloignent tellement du budget que nous avons votée fin 2020 et même après la maudit les modifications des Budgets rectificatifs, que c'est la portée même de l'autorisation parlementaire qui est en question, la Cour des comptes va même jusqu'à qualifier cette autorisation parlementaire, je la cite 2 malmené alors entre sous-exécution annulations et reports de crédits, notamment sur le plan de relance ce projet de loi témoigne de l'absence d'un pilotage rigoureux et efficace puisque les reports de 2020 sur 2021 était déjà d'une ampleur historique, mais en 2021 à nouveau les reports dépasse les 22 milliards d'euros et suivant des méthodes qui piétine les principes d'Amiens d'annualité et de spécialités budgétaire, cela a été dit par plusieurs collègues enfin sur le fond de la politique menée, nous aussi, nous regrettons que vous ayez laissé filer à ce point le déficit certes les indicateurs se trouve en 2021 améliorer sans qu'on puisse véritablement maître ce surcroît de recettes fiscales au crédit de la politique de gouverne du gouvernement, si ce n'est de ces hypothèses particulièrement particulièrement prudentes pour 2021, comme l'a noté la Cour des comptes, le gouvernement et d'ailleurs un peu piégé par sa propre contradiction qui consiste à mélanger dans son discours auto-satisfecit et à l'arme sur la côte d'alerte. Face à l'accroissement du déficit et de la dette de l'État, la majorité sénatoriale vous reproche elle de ne pas suffisamment maîtriser les dépenses sont toujours dire lesquelles, avouons-le, c'est largement vrai mais cette non-maîtrise ne vous conduit pas non plus à dégager des marges de manoeuvre pour une politique ambitieuse, que ce soit face à l'urgence sociale face aux nécessités de la transition énergétique ou pour remettre à niveau les services publics et surtout vous restez arc-bouté sur votre politique de l'offre prise prive l'État de ressources en même temps qu'elle accroît les inégalités, beaucoup a déjà été dit sur le ruissellement et ses illusions, rien ne prouve que la politique de l'offre à diminué à dynamiser la croissance mais c'est certain qu'elle a dégradé les finances publiques et entraver les marges de manoeuvre qui vous font tant défaut aujourd'hui, alors Monsieur le Ministre je conclurai par une question : en matière de politique de l'offre, c'est-à-dire de baisse d'impôts pour les entreprises et ceux qui détiennent les plus gros patrimoines allez-vous également passer du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte ce que Pascal Salvodelli a appelé le qui va payer. Je pose la question et comptez sur nous pour faire dès le projet de loi de finances rectificative des propositions concrètes en ce sens, je vous remercie. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, l'examen de la loi de règlement dans une entreprise, c'est un moment décisif, c'est le bilan, c'est l'instant de vérité dans le monde économique et normalement, ça a été souligné ça devrait être le cas pour l'État exemplaire et notamment dans les relations entre l'exécutif et le Parlement, malheureusement, nombreux ont été les orateurs qui ont souligné monsieur le Ministre ce dysfonctionnement initial dans le gouvernement, où vous faites partie et on peut vraiment se demander quelles sont les raisons de ce dysfonctionnement est-ce véritablement de l'impréparation de la part de Bercy ce serait surprenant mais ce serait une première S de la désinvolture au moment où, au contraire, on explique qu'on aime tout le monde, on aime les institutions et caetera c'est surprenant est-ce un sentiment de panique ce que par hasard, ce ne serait pas tout simplement le moment où on veut éviter une rencontre et notamment une rencontrent parce que dans la république, on vit un instant décisif, celle où un gouvernement se succède à lui-même et on a une loi de règlement qui va pouvoir faire le bilan de la loi de programmation des finances du premier quinquennat. En septembre 2017, le ministre des Finances a annoncé que l'objectif de cette loi de programmation c'était suppression des déficits ou abaissement des déficits abaissement des dépenses et abaissement des prélèvements obligatoires, alors inutile de dire qu'effectivement il y a toujours des événements, mais vous avez tout faux, ou en tout cas le quinquennat précédent le gouvernement précédent a tout faux et il y a un problème alors pour ma part, je m'arrêterai sur deux 3 choses parce que beaucoup de sujets ont été évoqués, mais ce qui m'intéresse moi, c'est les prélèvements obligatoires et sur les prélèvements obligatoires en dehors de l'année 2019, vous avez toujours fait mieux que sous le quinquennat de François Hollande, c'est une constatation, c'est une réalité, ils ont toujours été supérieurs que sous le quinquennat de François Hollande, il y a une sorte de continuité entre le quinquennat du président Macron et du président Hollande c'est un choix politique, en tout cas c'est ma vision des choses, et donc sur ce plan là, je pense que on est dans la continuité d'une certaine politique social-démocrate, c'est un choix, vous devez l'assumer, mais c'est quand même une réalité, ce n'était pas l'objectif initial que vous vous étiez fixé, c'est pour ça qu'il y avait une certaine séduction vis-à-vis des classes économiques vis-à-vis du monde de l'entreprise, mais lorsqu'on fait le bilan de cette loi de règlement, on voit que vous êtes à côté de la plaque en réalité vous n'y êtes pas arrivé et ça c'est un constat et c'est embêtant parce que les prélèvements obligatoires, c'est le pouvoir d'achat, alors vous êtes obligés à la vite de faire une loi sur le pouvoir d'achat, mais c'était simple : si vous aviez tenu vos engagements, pas vous, Monsieur le Ministre, mais le gouvernement précédent et l'objet du président de la République, il ne serait pas nécessaire peut-être malgré la crise, de faire une loi sur le pouvoir d'achat parce que la réalité, elle est là, dans ce pays, le pays d'Europe où avec l'Autriche, on est obligé de travailler plus de la moitié de l'année pour payer les services publics, payer l'État payer des collectivités territoriales, la protection sociale, c'est la réalité, ça n'a pas baissé, vous savez comme moi que c'était le 17 juillet il y a quelques jours, le jour de ce qu'on appelle la libération fiscale puisque, pour un entrepreneur, il faut mettre 220 euros pour que finalement un salarié un collaborateur puissent avoir cent euros de pouvoir d'achat 20 pour 100 de plus que tous les autres pays de l'Union européenne, pratiquement malgré tout, le bilan que vous avez tenté d'exposer, je dirais presque avec la tonalité d'un porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire quelqu'un qui sait bien communiquer et et faire montrer le bon côté des choses, la réalité elle est là, il y a pas de pouvoir d'achat, il y a des difficultés, il y a 9 millions de Français qui ont des difficultés à vivre et qui sont sous des seuils critiques et c'est ça le réel bilan de votre loi de règlement alors sur les dépenses, on prend l'exemple de la crise, mais c'est la Cour des comptes, c'est pas nous qui dit les dépenses non liées à la crise du Covid ont augmenté de 5,7 virgule je me souviens plus c'est quand même un, un bilan très lourd à porter, alors vous prenez vos fonctions, mon collègue Bachere là dit avec beaucoup de talent, jusqu'au 17 juillet le citoyen et les entreprises travaillent pour l'État. Et puis, à partir du mois d'août ben l'état prend de la dette pour les générations futures pour boucler son budget, puisque grosso modo on on pourrait revoir les comptes, mais c'est à peu près 50 50 ou 60 40, on doit payer les services de l'État de notre État, à 40 % au mois près de 49 % avec la dette, c'est ça la réalité d'un Français aujourd'hui par cette loi de règlement qui fait le bilan, le constat de 5 années d'un plan qui dorment allemande été idyllique pour nos finances publiques, alors les besoins de financement c'est évidemment dramatique parce que ce que je n'ai pas entendu dans les propos, ce sont des propos concernant l'avenir, pourtant, vous avez un âge où vous devrez parler aux générations futures la transition énergétique, ça été évoqué tout à l'heure, je crois que les besoins de l'Europe, c'est 350 milliards qui sont prévus d'ici quelques années, il y a l'investissement dans le numérique ou si on en parle beaucoup mais on est à la traîne derrière la, derrière les États-Unis, on est en retard en recherche et développement, ce sont quand même des sujets qui impacte nos sociétés pour l'avenir, je parle pas évidemment de l'énergie du militaire de la crise internationale, donc en réalité lorsque je suis rentré au Parlement, on ne votez jamais contre une loi de règlement, ça n'existait pas, ont considéré que comme dans un certain nombre de Budgets régaliens c'était porter atteinte à l'image de la France qui a emprunté sur les marchés internationaux et c'était très difficile, c'était des circonstances exceptionnelles et malheureusement la dégradation ces dernières années de nos finances publiques sous l'autorité des gouvernements qui se sont succédé, fait que pour la deuxième fois, je crois, ou la 3ème fois nous sommes obligés dans sont enceintes, tous partis confondus, pratiquement tous groupes politiques confondus, de voter contre cette loi de règlement, alors évidemment, pas de chance pour vous, Monsieur le Ministre, vous prenez vos fonctions pour un baptême du feu, on pourrait dire que c'est un petit peu délicat, mais il y a presque unanimité l'unanimité, ça me permet de revenir sur mon propos initial est ce qu'il n'y avait pas un peu de panique. Dans ce retard, faut pas revenir

Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues. La loi de règlement, c'est le moment de vérité. Je regrette cette année encore, que nous n'y consacrions pas davantage de temps. Cela nous permettrait de remplir pleinement la mission d'évaluation et de contrôle qui nous incombe. L'exercice 2021 et le dernier du quinquennat. Il est l'occasion de dresser le bilan de la gestion financière de l'exécutif. 170 milliards de déficit en 2021, la France enregistre le pire niveau de son histoire après 2020.

Notre dette atteindra prochainement 3000 milliards, c'est-à-dire 10 ans de recettes d'impôt, impôt sur le revenu un peu sur les sociétés, TVA. à ce niveau, si les taux continuent de remonter, imaginons qu'ils atteignent 5 % c'est pas totalement impossible, non, non, mais c'est peut-être beaucoup, mais c'est peut-être pas totalement impossible, ça fait combien ça fait, ça fait 150 milliards de coût annuel, voilà ce que ça coûte la dette ça peut coûter 150 milliards, c'est-à-dire 2 fois le budget de l'Éducation nationale. C'est colossal, déjà en 2022, Bercy prévoit de verser 55 milliards au marché qui nous financent et ceux qui haïssent ces marchés financiers, il y en a quelques-uns sont les mêmes qui voudrait leur en donner davantage. Cessons le feu, il est grand temps de revenir à une gestion rigoureuse et sérieuse, notre argent public. La dérive de nos finances publiques est antérieure à l'apparition du virus. Les dépenses courantes, sans lien avec la crise sanitaire ou la relance économique auront augmenté de près de 140 milliards sur la durée du quinquennat. Pire, le déficit structurel a doublé en l'espace de 5 ans, passant de 72 à 145 milliards d'euros. Le contexte favorable des 3 premières années du quinquennat aurait dû être mise à profit pour assainir nos comptes publics et désendetter le pays. Non seulement le niveau d'alerte est atteint, mais il est largement dépassé, la faute à une absence totale d'ambition et 100 matrice. Et a après. Alors que faire. Tout d'abord sortir du groupe des pays dits du Club Med et prendre exemple sur les pays sérieux en matière budgétaire et Lyon. Mais aussi prendre exemple sur les collectivités territoriales, monsieur le Ministre, certes, rares sont les ministres à avoir été à la tête d'un exécutif local, et c'est bien dommage, mais cela ne devrait pas priver l'État de suivre leur saines pratiques en matière de gestion des finances publiques. Depuis 2017, à l'exception de 2021, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont toujours connu une croissance égale ou inférieure à l'inflation. Or, si l'État s'en était lui aussi tenu à l'inflation, ces dépenses auraient été en 2021 inférieur de 50 milliards d'euros CAC sur le quinquennat nous aurions 210 milliards de dettes de moins. Alors que l'État Zakopane à empiler les déficits budgétaires pendant 5 ans, les collectivités locales, elles ont toujours enregistré un solde excédentaire, exception faite de l'année 2021 où il ne s'est toutefois dégradée que de 600 millions d'euros à rapprocher avec les 170 milliards de déficit de l'État. C'est que les élus locaux, contrairement aux décideurs de l'État sont astreint à respecter une règle d'or, les enjoignant à respecter l'équilibre du fonctionnement et à ne procéder à l'emprunt que pour l'investissement. Il y a urgence à contraindre à l'identique les finances de l'État. Monsieur le Ministre, il va vous falloir du courage, du courage et encore du courage. Pour rétablir les grands équilibres du budgétaire si c'est le cas, nous serons à vos côtés pour vous aider à prendre les décisions qui s'imposent, ce qui m'inquiète, c'est que visiblement ne l'avons pas la même conception de comptes bien tenus et de la vertu en matière de finances publiques. Le groupe Union centriste essaiera lors du prochain PLFR de vous montrer la bonne voie pour être sur une dynamique vertueuse en la matière, je vous remercie. Merci. La discussion générale étant Close, nous allons passer à la discussion des articles du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale Oui merci madame la présidente, c'était simplement pour répondre à la discussion générale, je veux remercier d'abord l'ensemble des Z'orateurs qui se sont exprimés remercier chacune et chacun des sénateurs qui sont présents et sont restés pour ma réponse, je vais revenir le plus et madame derrière le plus exhaustif possible sur sur les différents sujets qui ont été évoquées, même si dans beaucoup des interventions, on voit bien que les débats que nous aurons prochainement sur le projet de loi de finances rectificative sur le projet de loi de finances pour 2023 sur la loi de programmation pour les finances publiques seront nourris et seront très très nombreux, je veux d'abord revenir sur cette question du calendrier. Oui, c'est important, le calendrier, c'est important de donner au Parlement, la possibilité de travailler sur les textes en amont de leur discussion et j'ai le plus grand respect pour nos règles et pour évidemment la loi organique, vous avez semblé présentée comme une grande première, le fait que ce projet de loi de règlement a été présenté, après le délai prévu et la date prévue par la loi organique, j'ai été regardé dans les années précédentes, ou plutôt les quinquennats précédents, ce qui s'était passé à la première année de chacun des quinquennat il s'est assez strictement la même chose que cette année. C'est-à-dire une présentation du projet de loi de règlement au 1er, conseil des ministres, qui fait suite aux élections législatives, c'est exactement ce qui s'est passé en 2017 quand Emmanuel Macron a été élu la première fois, c'était ce qui s'était passé Monsieur Féraud en 2012 quand François Hollande a été élu, projet de loi de règlement présenté après le délai de la loi organique, c'était ce qui s'était passé en 2007, quand Nicolas Sarkozy avait été élu, projet de loi de règlement présenté après le délai de la loi organique après les élections législatives, il s'agit pas de dire que, on l'a présenté, après le délai de la loi organique parce que ça a toujours été fait comme ça, il y a des raisons, il y a eu des élections législatives le déposer avant aurait impliqué de redéposer une deuxième fois le même texte et de faire de dépôts puisque l'Assemblée nationale a été renouvelé au moment des élections législatives et surtout nous avons voulu voulu tenir compte dans le projet de loi de règlement de la croissance constatée par l'Insee en 2021 dont les indicateurs nous ont été communiqués au 31 mai, raison pour laquelle nous avons déposé le projet de loi après cette date, mais je le dis de manière très claire, nous respecterons dans les années qui viennent, le délai qui est prévu par la loi organique, y compris après révision de la loi organique par la PPL au Woerth Saint-Martin dont vous avez parlé, qui prévoit d'avancer, je crois au premier mai le délai de dépôt pour le projet de loi règlement ce sera tenu, mais encore une fois, je veux vraiment démentir cette idée que ce serait une grande première en allait électorale que le projet de loi est déposée après le délai de l'organique, ça a été le cas strictement à chacune des années électorales, je veux revenir sur d'autres sujets transversaux qui ont été évoqués par plusieurs d'entre vous, notamment sur la question des reports de crédits que vous avez qualifié d'exceptionnel, c'est vrai qu'ils ont été explique notamment en 2020 pour l'année 2021, un peu moins pour l'année 2021 pour l'année 22, vous avez en tout cas un certain nombre d'orateurs omis de dire qu'il s'agissait d'année exceptionnelle. Et que quand vous faites face à une crise telle que celle que nous avons connu avec la crise sanitaire, oui, cela implique de prévoir des Budgets dans un contexte d'incertitude et il vaut mieux prévoir entre guillemets à grosses mailles pour ne jamais être en rupture de paiement, plutôt que de se retrouver dans une situation, on n'est pas capable de payer pour des tests ou pour des masques parce qu'on n'a pas prévu assez je veux quand même indiqué que nous avions avant cette année exceptionnelle de la crise sanitaire remis de l'ordre dans cette question des reports. On s'était d'ailleurs engagée en 2017 avant l'élection d'Emmanuel Macron, en 2017, le volume des reports de crédits d'une année sur l'autre était autour de 3 milliards d'euros pour 2016 à 2017, c'était 3 milliards 500 millions d'euros, 2017 à 2 1000 18 premières années donc du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, 1,7 milliard 2018 à 2019, 2 milliards, on reste dans ces ordres-là 2019 à 2020, 1 virgule 9 milliards, donc on a vu dans les 3 premières années du précédent quinquennat que nous avions très largement réduit le volume des reports d'une année sur l'autre, il y a eu davantage de report au moment de la crise sanitaire, je l'admets volontiers, je le constate, ils ont été réduits l'année dernière et nous les réduirons encore une fois cette année, pour continuer à tendre vers cet objectif du plus faible niveau de report possible sur ensuite les résultats que vous avez qualifié de moins bon que nos voisins, moi je veux quand même rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, la France est le 1er le seul pays de la zone Euro, avoir retrouvé son niveau économique d'avant crise au 3ème trimestre 2021 dès le 3ème trimestre 2021, vous nous avez comparé à nos voisins.

pour l'Italie, plus 0 5 pour 100 pour l'Espagne, moins de 3 % donc nous allons plus vite que la plupart de nos voisins dans le rétablissement de notre site, notre activité économique et nous avons retrouvé notre niveau d'activité économique pré-crise avant nos grands voisins c'est à saluer, mais indépendamment de l'action du gouvernement, il faut saluer l'ensemble des entrepreneurs, l'ensemble des entreprises, ensemble des salariés. Qui se sont mobilisés pour nous permettre de rebondir aussi rapidement Madame briquet, vous avez évoqué la question du solde structurel, oui, il y a une dégradation affiché du solde structurel dans ce projet de loi de règlement pour une raison, entre guillemets, simple, c'est que des dispositifs qui étaient qualifiés ou qui étaient comptés comme des dispositifs temporaires en 2020, notamment liés à la crise économique liée à la crise sanitaire, je pense au fonds de solidarité à l'activité partielle ont été qualifiés en 2021 comme dispositif structurel parce que c'est de la sincérisation budgétaire ils ont duré plus longtemps qu'une année, ce qui était prévu au départ, ce qui explique la dégradation légère de notre solde structurel mais cette dégradation est temporaire, puisque ces dispositifs ont vocation à s'éteindre quand ils ne se sont pas déjà éteint en 2022 puisque nous ne sommes plus dans la même dans je veux revenir sur un certain nombre de questions qui ont été posés en tout cas de critiques qui ont été émises sur la stratégie budgétaire, fiscale et économique du gouvernement, je pense à Monsieur Savoldelli à Monsieur Féraud, par exemple, qui ont critiqué notre choix effectivement de baisser les impôts, ce qui répond en fait quelque part à monsieur Dominati, qui estimait que nous n'avions pas baisser les impôts et que nous avions une forme de continuité avec le quinquennat précédent, celui d'Emmanuel Macron sur ce sujet là, non, les impôts n'ont pas baissé de 50 milliards d'euros dans le quinquennat de François Hollande, contrairement à celui d'Emmanuel Macron je le sais, j'y étais. Nous avons baissé les impôts de 50 milliards d'euros avec Emmanuel Macron 25 milliards pour les ménages, 25 milliards pour les entreprises et nous allons continuer à le faire, ça a d'ailleurs été non pas saluer, mais en tout cas, notez par les sénateurs, ça vous le délit et Ferrero je veux simplement dire que, quand bien même nous avons baissé les impôts, nous collectons davantage. La l'impôt sur les sociétés, son taux est passé de 33 % à 25 % et pourtant l'an dernier, nous avons collecté davantage en volume à un taux de 25 % que ce que nous collections à 33 %, c'est ce qui a été souligné notamment par le sénateur Rambo dans son intervention, le sénateur qui a pu également, ça montre bien que nos stratégies de faire baisser la pression fiscale sur nos entreprises pour favoriser l'activité économique est une stratégie payante ensuite d'abord d'un point de vue économique mais aussi d'un point de vue des finances publiques puisque nous collectons davantage de recettes baisser les impôts baisser le coût du travail, ça favorise l'activité économique et l'emploi, plus vous favoriser l'emploi plus, ce sont aussi des recettes pour la puissance publique. Financer nos services publics et notre modèle social puisque plus il y a de Français qui travaillent, plus il y a de cotisations qui sont versés, moins il y a d'indemnisation chômage qui est versée, et donc c'est bon pour les finances publiques aussi et ça les chiffres en en en attestent, monsieur Beuchere, j'ai bien entendu l'ensemble de votre intervention, vous êtes, vous êtes vous êtes redescendu je veux d'abord vous rassurer sur la question du calendrier du report, le programme de stabilité sera présenté très prochainement, avant la fin du mois, oui, nous avons demandé à la Commission européenne, comme ça se fait régulièrement au moment des élections pour d'autres pays que la France y compris de pouvoir présenter notre programme de stabilité plus tard et la Commission ne s'y est pas opposé et je pense qu'on nous aurait critiqué si on avait présenté un programme de stabilité juste avant les élections présidentielles, on nous aurait dit vous engager la France sur une trajectoire avant un moment démocratique majeur, vous devriez attendent les élections présidentielles pour que la nouvelle majorité, le nouveau gouvernement construisent un programme de stabilité donc il sera présenté avant la fin du mois, ce sera l'occasion de débattre ensemble de débattre au Parlement, je veux simplement revenir sur les questions de gestion budgétaire que vous avez évoquée de dérapage des finances publiques, je sais parfaitement que je suis au Sénat et que chacun des groupes parlementaires entre l'Assemblée nationale et le Sénat sont autonomes, mais je crois quand même à l'existence de formation politique, il se trouve que nous examinons cette semaine le projet de loi de finances rectificative pour 2022, à l'Assemblée nationale et que le délai de dépôt des amendements pour la première lecture s'est arrêté hier à 17 heures que j'ai été regarder les amendements du groupe, les républicains à l'Assemblée nationale sur 447 amendements. Il n'y a que des amendements de dépenses supplémentaires ou de moindres recettes pour un montant global de 100 milliards d'euros, 100 milliards d'euros sur ces 447 amendements, il n'y en a que 25 qui ne prévoit pas des dépenses supplémentaires ou des moindres recettes, ce sont 25 demandes de rapport, je pense que c'est pour plaire au Sénat aussi, mais en tout cas, voilà, je veux dire moi je, j'entends parfaitement les leçons et on est, je suis aussi là pour les écouter, pour échanger, mais encore faut-il. Faire preuve de sérieux budgétaire dans les propositions que l'on n'aimait et dans les amendements que l'on dépose mais je suis sûr que lors de l'examen de ce texte par le Sénat, cet été, ce sera autre chose, et les dépenses nouvelles qui seront proposées ou demander seront financés par des réformes de structure puisque c'est ce que vous appelez de vos voeux, je veux revenir sur quelques questions plus particulière qui ont été posées, Bruyère sur la question des ETP supprimés au ministère de la transition écologique, en réalité, il y a 2 effets majeurs en 2021 et notamment un effet dis ce puisqu'il y a un certain nombre d'effectifs qui ont été transférés entre administrations ne relevant pas nécessairement du même ministère avec un changement d'organisation interne, notamment dans le cadre de la création des secrétariats généraux des directions départementales interministérielles, c'est principalement en effet de périmètre, il y a aussi un effet de schéma d'emplois du ministère où effectivement il y a depuis plusieurs années un peu plus de recrutement d'agents de catégorie à une réduction des agents de catégorie, c'est ce qui explique une partie de la baisse du nombre de TP, mais en tout cas, il y a aussi cet effet périmètre dont il faut tenir compte pour expliquer ce volume de 2000 TP qui de 2000 TP qui sont, qui sont supprimés, monsieur Villach, vous avez évoqué la question de la situation des collectivités locales, là aussi, je pense que nous aurons l'occasion d'en parler ici, il y avait une réunion importante qui s'est tenue aujourd'hui avec mes collègues caille et Béchu. Avec les associations d'élus, précisément pour faire le point avec eux, on voit aujourd'hui une situation au global, je dis bien au global plutôt bonne pour les collectivités locales. épargne nette en très forte augmentation par rapport à 2019 plus 9 % des recettes réelles de fonctionnement qui augmente très fortement depuis le début de l'année sur les 5 premiers mois de l'année, c'est près de 5 milliards de recettes réelles de fonctionnement en plus pour les collectivités locales par rapport aux 5 premiers mois de 2021 pour autant, on sait qu'il y a certaines collectivités qui connaissent des difficultés, notamment en raison de l'inflation et nous aurons probablement dans les prochains textes. L'occasion d'échanger sur le meilleur moyen de venir les les soutenir, je crois que j'ai répondu à la majorité des questions en tout cas qui sont revenus régulièrement je terminerai en disant puisque vous avez dit monsieur Huchon, monsieur le rapporteur général que vous votiez contre ce projet de loi de règlement par cohérence avec le fait que vous avez voté contre la loi de finances. Initial que moi je j'ai toujours du mal à comprendre finalement pourquoi votent contre un projet de loi de règlement qui ne fait que prendre acte de ce qui s'est passé l'année précédente, je suis conseiller municipal dans ma commune depuis 8 ans, je vois très bien qu'on peut voter contre un budget quand on est dans l'opposition et voter pour le compte administratif, précisément parce qu'on regarde la photographie de ce qui s'est passé l'année précédente, on ne peut pas changer le passé. On peut le commenter, on peut en débattre, oh pas le changer, en revanche on peut construire l'avenir et je sais que c'est ce que nous ferons ensemble dans les prochains mois et je m'en réjouis. je vais donc nous passons donc maintenant aux articles je mets aux voix l'article liminaire avant l'article inquiet pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté à l'article 1er, une demande de parole de monsieur tant la Mini, vous avez la parole. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, concernant cet article, enfin tous les articles sont importants, j'interviendrai modestement sur cet article 1 qui correspond au résultat budgétaire de l'État en 2021 arrêtées à moins 170 7 milliards d'euros, s'agissant des recettes le montant Net des recettes hors fonds de concours s'élève à 316 milliards d'euros environ et à déduire, je crois que c'est important de le rappeler des collègues sont intervenus, notamment sur le volet collectivités territoriales, qui est aussi fondamentale, il y a un prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne, qui s'élèvent néanmoins 69 milliards d'euros, les recettes fiscales nettes augmente de 15,5 % par rapport à 2020 et s'élève à 295 milliards d'euros, a noté une baisse significative de la TVA à hauteur faire qui s'élève à 95 5 milliards pour l'année 2021 écoulé pour mémoire la TVA représenter 156 milliards d'euros en 2018 et c'est lié au transfert collectivités en direction des collectivités territoriales et des administrations de Sécurité sociale, s'agissant des des dépenses en crédits de paiement le s'élève à 557 milliards d'euros avec des missions importantes anciennement scolaire 75 milliards d'euros, la défense 49 milliards les engagements financiers notamment 38 4 milliards, donc s'agissant de cet article 1er néanmoins, à titre personnel, je m'abstiendrai. Merci, je mets donc aux voix l'article. Qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté à l'article de Monsieur la mini-vous souhaitez encore vous exprimer, je vous avez la parole. Alors s'agissant de de l'article de bons qui correspond au montant définitif de ressources et Charles de trésorerie qui ont concouru à l'équilibre financier, le besoin de financement, comme ça été rappelé s'élève à 285 milliards d'euros environ, dont le déficit a financé à hauteur de 170 milliards d'euros d'euros et l'amortissement de la dette notamment à moyen et long terme, à hauteur de 118 3 milliards d'euros à noter que la principale ressource, c'est l'émission de nouvelles dettes à moyen et long terme, à hauteur de 260 milliards d'euros en 2021 ans en reconnaissons que tout est particulièrement technique et en remercions, bien entendu, le rapporteur général et la commune, le président de la commission des finances, et tous les services pour aussi tout le travail d'expertise qui a été fait mais néanmoins je ne suivrai pas à titre personnel, l'avis de la commission et m'abstiendrai sur cet article également. Merci, je mets donc aux voix cet article 2 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, je me vois l'article 3 qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient qui n'est pas adopté, je me vois l'article IV qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté article 5 même vote il n'est pas adopté article VI même vote il n'est pas adopté article cette même vote il n'est pas adopté, mes chers collègues, nous en arrivons donc à l'article 8 je vous rappelle que si cet article n'était pas d'adopter, il n'y aurait pas lieu de voter sur l'ensemble du projet de loi dans la mesure où tous les articles qui le composent, auraient été supprimé en application de l'article 59 du règlement, le scrutin public et de droit sur l'ensemble du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des condamnés 2021, en conséquence, l'article 8 va être mis aux voix par scrutin public, quelqu'un demande si la parole pour expliquer son vote aux exprimer sur l'ensemble du projet de loi, je ne vois pas de demandes de parole je mets donc aux voix cet article par scrutin public qui va être ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert.

C'est bon, plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos. 343 exprimés 292 pour 57 contre 235 l'article 8 a donc pas été adopté les articles du projet de loi ont été successivement supprimé par le Sénat, je constate que sur l'ensemble du texte il n'aident pas donc pas nécessaire qu'il y a un vote en conséquence, le projet de loi n'est pas adopté, mes chers collègues, je vais lever la séance, la prochaine séance aura lieu mercredi 20 juillet à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement et la séance est levée.